Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le gouvernement nous demande d'avancer le début de l'examen du projet de loi, accélération de la production d'énergie renouvelable qui était initialement prévu jeudi 3. nous le l'avance serions le mercredi 2 novembre sans doute dans l'après-midi, à l'issue de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques 2023 2027 tu et données de cette demande. Nous pourrions fixer si vous en êtes d'accord, le délai 10 minutes d'inscription des orateurs dans la dire, déclare la discussion générale de ce projet de loi donc énergies renouvelables ou lundi 31 octobre à 15 heures et ce qu'il y a des observations. il est ainsi, il en est ainsi décidé et lors du jour appelle la discussion de la proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques présentée par Madame Éliane Assassi monsieur Arnaud Bazin et plusieurs de leurs collègues. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au vu de l'heure de reprise de nos travaux. Et en accord avec la Commission et le gouvernement, je vous propose d'ouvrir la nuit pour cette séance en nous assurant d'aller au terme de la discussion de ce texte. ça peut être évidemment un plus tard. Mais il me semble que c'est une position qui est largement partagée. Pas d'objection, il en est ainsi décidé. Et, bien entendu, chacun en tirera la conséquences en mettant le maximum d'intensité dans l'expression de ses opinions et réflexion dans la discussion générale, la parole revient d'abord à la présidente : Éliane Assassi, auteur de la proposition de loi. Pour dix minutes. Monsieur le président. Monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues, j'ai donc l'honneur de vous présenter notre proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil dans les politiques publiques, ce texte est le résultat d'un travail rigoureux de la commission d'enquête du Sénat, créé à l'initiative de mon groupe, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, il s'appuie sur 4 mois d'investigations, 40 auditions et l'analyse de 7300 documents, nous poursuivons trois objectif : en finir avec l'opacité des prestations de conseil mieux les encadrer et renforcer les exigences déontologiques des consultants, il ne s'agit pas là d'interdire par principe le recours aux cabinets de conseil, mais bien de fixer un cadre clair pour mettre fin aux dérives constatées par la commission d'enquête cette démarche transpartisane elle associer tous les groupes politiques de notre assemblée, je veux ici remercier l'ensemble des membres de la commission d'enquête pour leur soutien, ainsi que la commission des lois, et sa rapporteure Cécile Cukierman pour les améliorations apportées au texte, c'est le pluralisme sénatorial qui s'exprime ce soir, je crois que nous pouvons en être fiers, sur tous les bancs de notre hémicycle je souhaite également remercier très sincèrement le président Arnaud Bazin qui était fut également président de la commission d'enquête avec qui nous travaillons de concert dès le 1er jour, la commission d'enquête a mis au jour un phénomène tentaculaire, l'influence croissante de consultants privés sur des pans entiers des politiques publiques, la crise sanitaire, la stratégie nationale de santé, l'avenir du métier d'enseignant, la mise en oeuvre de la réforme des APL, les états généraux de la justice, la liste des missions déléguées à des cabinets privés et tellement foisonnante qu'elle en donne le tournis au point de se demander si il y a un pilote dans l'avion, en 2021, la facture des consultants s'élève à au moins 1 milliard d'euros pour l'État et ses opérateurs, elle a plus que doublé depuis 2018, en pratique, les cabinets conseils n'ont pas de problème de pouvoir d'achat. Une journée de consultants coûte en moyenne 1500 euros à l'État, ce chiffre ayant atteint 2168 euros pendant la crise sanitaire malgré ce niveau de rémunération, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Cap Gémini a par exemple reçu de 180200 euros pour une mission sur le handicap, alors que l'évaluation parle, je cite, d'une valeur ajoutée quasi nulle parle du cabinet bien évidemment contre- productif, parfois, BCG et Ernst and Young ont reçu 558900 euros pour organiser une convention des managers de l'état en décembre 2018 qui n'aura finalement jamais lieu McKinsey a reçu en novembre 2019 9000 157000 euros pour une mission commandée par pour par la CNAV visant, je cite encore à aider la caisse à se transformer en vue de la réforme des retraites, alors que celle-ci, tout le monde s'en souvient, a été abandonné, de telles dérives sont inacceptables, surtout lorsqu'il s'agit d'argent public et surtout dans le contexte actuel, au quotidien, l'opacité règne sur les prestations des cabinets de conseil, qui souhaite rester excusez l'anglicisme behind pour reprendre leur expression à titre d'exemple, la Commission Cyrulnik sur les 1000 premiers jours de l'enfant n'était pas au courant que l'État avait missionné le cabinet Roland Berger en parallèle de ces travaux, ce cabinet a touché plus de 420000 425000 euros pour un travail qui, je ne suis je cite encore, n'était pas à la hauteur d'un cabinet de stratégie selon donc l'évaluation de la DTP dans le même temps, les membres de la commission Cyrulnik, médecin expert de haut niveau était bénévole et avait du mal à se faire rembourser leurs frais de déplacement pour se rendre aux réunions, c'était 2 poids 2 mesures, si notre commission d'enquête a été un exercice de transparence démocratique, on constate un retour à l'opacité depuis au-delà de l'exercice de communication, le jaune, que le gouvernement a publié la semaine dernière et là qu'une aire et je dois dire très décevant lacunaire car il exclut le conseil en informatique et ne couvre que la moitié du périmètre de la commission d'enquête, il ne concerne que 470 millions d'euros de prestations contre 894 millions dans nos travaux, les chiffres parlent d'eux-mêmes, décevant car le gouvernement se refuse à publier la liste de ses prestations de conseil alors qu'il s'agit d'une information essentielle, que nos concitoyens sont en droit de connaître, en pratique, les ministères, traîne des pieds pour répondre aux demandes des journalistes, entretenant ainsi ce climat d'opacité pour gagner du temps, l'État refuse toujours de communiquer des documents malgré les avis, les avis favorable de la Cada, le 21 janvier dernier, un journaliste de Next Inpact demandait au ministère de l'Éducation nationale, une copie du rapport de McKinsey sur l'avenir du métier d'enseignant facturé pour une somme exorbitante de 496800 euros 10 mois plus tard, il attend toujours le 12 octobre le journal Le Monde annoncé sa volonté de saisir la justice face aux non-réponse de l'Élysée, de Matignon et de la plupart des ministères, le gouvernement ne doit pas avoir peur de la transparence, bien au contraire, c'est pourquoi notre PPL imposera la publication de la liste des prestations de conseil de l'État et de ses opérateurs ainsi que des bons de commande et des évaluations de prestations ces informations figureront dans le rapport social unique pour que les fonctionnaires puissent en débattre les agents publics ressentent en effet un profond malaise lorsque des consultants viennent leur expliquer leur métier à coups de post-it de jeux de rôles ou encore de Paper board, c'est le cas à l'Ofpra ou les consultants de Wavestone chasse ce qu'ils appellent des irritants pour réduire le délai de traitement des demandes d'asile autre exemple pendant la campagne de vaccination McKinsey utilisant le logo de l'administration pour rédiger ses livrables Véran, ancien ministre de la Santé d'affirmer devant notre commission d'enquête, je cite encore : si vous aviez voulu les documents estampillés McKinsey, présent dans le dossier, vous auriez trouvé une feuille blanche, c'est étrange pour une prestation facturée plus de 12 millions d'euros, c'est pourquoi nous souhaitons éviter toute confusion entre les fonctionnaires et les cabinets de conseil qui ne qui ne pourront plus utiliser les signes distinctifs de l'administration, à l'initiative de Michael Valette, nous proposons de bannir les expressions anglo-saxonne d'inspiration managérial comme benchmark lean management ou encore que leur nid, conformément à l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français, y compris pour les consultants, certains ont résumé notre texte à la PPL dites McKinsey certes les pratiques de ce cabinet ont choqué nos compatriotes en particulier sur le plan fiscal 0 impôt sur les sociétés pendant 10 ans, alors que son chiffre d'affaires atteint 450 millions par an, comble de l'ironie, le 11 juillet dernier sur BFM Business, la directrice générale de McKinsey rejeter la faute sur le coût du travail en France qui reste bien évidemment trop élevé à son goût, en réalité, McKinsey peut remercier le mécanisme des prix de transfert et le paradis fiscal du de l'ovaire, il continue d'ailleurs de candidater au marché public, il a été désigné titulaire de son courant du marché de l'UGAP attribué en plein été, mais notre proposition de loi va bien au-delà de ce seul cabinet le recours aux consultants est devenu un réflexe pour l'administration, alors qu'elle dispose des compétences en interne, on a parfois l'impression que l'État se fie davantage au PowerPoint de ces consultants qu'au travail de ces de le recours croissant au cabinet de conseil illustre une certaine vision de l'État, un État en mode Start-Up pour reprendre le titre d'un ouvrage évoqué pendant l'audition de McKinsey en déléguant ses missions stratégiques à des cabinets privés, l'État risque toutefois de perdre de perdre en souveraineté au bénéfices des multinationales du Conseil, nous serons tous d'accord pour éviter, a-t-elle risque le gouvernement lui-même a d'ores et déjà pris des mesures, la plupart du temps en réaction à nos travaux, nous gardons bien évidemment à l'esprit la circulaire signée le 19 janvier le 19 janvier dernier, le même jour, de l'audition d'Amélie de Montchalin devant notre commission d'enquête, le hasard fait parfois bien les choses, monsieur le Ministre, le gouvernement a besoin de notre PPL pour mieux encadrer le recours aux cabinets de conseil, vous le savez, car nous en avons, nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur le sujet de manière franche et directe, c'est pourquoi nous vous demandons solennellement d'inscrire notre proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, sans en réduire l'ambition, nous avons un devoir de responsabilité vis-à-vis des Français qui se sont emparés du sujet et qui souhaite que les choses changent, l'enjeu dépasse même notre pays le 30 septembre dernier Radio-Canada annoncé que McKinsey avait été payé 35000 dollars par jour pendant la crise sanitaire au Québec dans l'opacité la plus totale, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons ensemble le devoir de fixer des règles plus claires pour les consultants dans l'intérêt de l'État et de nos politiques publiques, ce n'est pas qu'un souhait des parlementaires que nous sommes dans notre diversité, c'est une exigence devenu populaire au fil des travaux de notre commission d'notre débat de ce soir est attendu et je fais confiance à notre Haute assemblée pour être à la hauteur de ses exigences, je vous remercie. La parole est à présent. Madame Cécile Cukierman, rapporteur de la commission des lois. Monsieur le président, monsieur le président de la commission de loi Monsieur le Ministre, pardon, mes chers collègues, la proposition de loi de nos collègues, Éliane Assassi Arnaud Bazin est ambitieuse et profondément novatrice, elle a été nourrie par les travaux que la commission d'enquête a conduit pendant plusieurs mois sur l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques, ces travaux ont suscité de nombreuses réactions du gouvernement et de l'administration comme des consultants circulaire du Premier Ministre refonte de l'accord-cadre de la Direction interministérielle de la transformation publique dont l'équipe de conseil interne doit être renforcée, rédaction par l'organisation professionnelle Syntec, conseil d'une charte de déontologie spécifique pour les interventions de conseil auprès du secteur public et très récemment publication par le gouvernement d'une annexe au projet de finances pour 2023, vous me permettrez monsieur Ministre de ne pas utiliser ici l'expression de jaune budgétaire mais je pense que nous irons viendront si ces initiatives vont dans la bonne direction, elle, reste insuffisante, n'ayant pas le caractère général et pérenne souhaité la commission des lois, estime par conséquent qu'une loi instituant un cadre unifié contrôler et sanctionner est aujourd'hui nécessaire, le texte proposé par nos collègues Éliane Assassi Arnaud Bazin répond à quatre ans, je tousse essentielle dans le cadre d'une démocratie que l'on souhaite mature, un enjeu de transparence vis-à-vis des parlementaires, mais surtout à destination des citoyens, un enjeu de maîtrise de la dépense publique, un enjeu de souveraineté à travers l'action de l'État, et enfin un enjeu de probité. Il a été co-signé par la quasi-intégralité des membres de la commission d'enquête est le fruit d'un travail transpartisan. La commission des lois a donc tenu à conserver cet équilibre tout en l'ajustant pour lui apporter une pleine effectivité dans cet esprit, elle a sécurisé le périmètre de la proposition de loi en choisissant une rédaction plus précise, juridiquement, préférant la catégorie des établissements publics de l'État à celle d'opérateur et en évitant les chevauchements de compétences avec les conseils de discipline des professions réglementées, de droit, elle a renforcé l'exigence de transparence et clarifier le partage des responsabilités entre administration et consultant, la commission a également rendu plus dissuasive, l'amende administrative qui seraient exigées des personnes morales ne respectant pas les nouvelles obligations mises en place en la portant à un montant proportionnel à leur chiffre d'affaires mondial, elle a enfin apporté des garanties à la procédure de vérification sur place et créer un mécanisme de régularisation en cas d'exclusion des procédures de passation des marchés publics, cela étant dit, j'ai bien conscience que le texte adopté par la commission n'est qu'un point d'étape et non un aboutissement certains sujets importants restent en effet en débat mais il nécessite le temps de la réflexion que permet la navette et le débat parlementaire, il en va ainsi du Champ d'application de la proposition de loi s'agissant aussi bien des administrations bénéficiaire que des prestations de conseil concernés pour ce qui est de la liste des administrations bénéficiaires tout d'abord la question de l'inclusion ou non des collectivités territoriales se pose, c'est indéniable, loin de nous, d'ailleurs l'idée d'opposer un État friands de prestations de conseil à des collectivités territoriales qui n'y recourait jamais toutefois, cette question ne peut être réglée sans consulter les associations d'élus locaux et sans comprendre quelles en seraient les conséquences sur le fonctionnement de ce même collectivité territoriale, nous n'allons donc pas le faire au détour d'un amendement de séance ce serait alors affaiblir, y compris les objectifs vous. De même, la question des seuils et récurrente, y compris pour les établissements publics de l'État que que nous avons intégré dans le Champ d'application de la proposition de loi, cependant, en l'absence d'informations permettant d'établir la liste précise des établissements publics concernés par telle ou telle seuil, il me semble prématuré à ce stade de en fixe de dans le même ordre d'idée, la liste des prestations de conseil entrant dans le Champ de la proposition de loi mériterait très certainement d'être affiné ultérieurement à ce stade, le gouvernement et quelques-uns de nos collègues ont donc formulé un certain nombre de propositions, une partie d'entre elles remettent en cause l'architecture du texte, en particulier le rôle accordé à la Haute autorité à la transparence de la vie publique et le recours à des sanctions administratives ou reviennent sur la substance des obligations mises à la charge de l'État, en particulier en matière de transparence, c'est pourquoi la Commission s'y opposera, d'autres suggèrent des modifications plus restreinte, nous ne les avons pas retenue à ce stade, pour nous concentrer sur le cadre général, nous pourrons pour certaines très certainement y revenir dans la suite de la navette enfin certains auraient souhaité saisir l'occasion de ce texte pour renforcer le cadre législatif s'appliquant aux représentants d'intérêts, ils en ont été empêchés par l'article de la par l'application de l'article 45 de la Constitution et surtout, là encore, la volonté de préserver l'équilibre de cette proposition de loi issus du travail de la commission d'enquête ce sujet demeure cependant important et mériterait un texte à part notre comité de déontologie mènent d'ailleurs une réflexion sur les règles applicables aux représentants d'intérêts au Sénat. Je crois que ce soir, nous fixons un cadre nous coulons en quelque sorte les fondations, mais tout ne sera pas terminé ce soir et après l'examen du texte ici au Sénat, il y aura besoin, comme je l'ai déjà dit de poursuivre le dialogue, d'améliorer, pour rendre applicable et effective, cette proposition de loi notre rôle ici n'est certainement pas d'affaiblir l'État et à travers, lire notre République, il est au contraire de chercher à prendre les meilleures décisions pour changer des pratiques qui ont conduit progressivement à externaliser une partie de la prise de décision vers le secteur privé, nous ne sommes donc pas là pour tout renverser, mais bien pour mener pleinement notre rôle de parlementaire, celui du travail de contrôle comme celui d'initiative législative et donc nous ne doutons pas que l'Assemblée nationale fera de même sera pleinement son rôle et inscrira et examinera dans les semaines, les mois à venir, cette proposition de loi pour conclure la commission vous invite donc à adopter son texte enrichi de quelques amendements pour poser comme je l'ai dit, les premiers grands jalons de l'encadrement de l'activité des cabinets de conseil auprès de l'État et de ses administrations dans un délai qui nous a été contraint par le temps, nous aurions certainement eu loisir de mener plus d'audition certainement plus longtemps, mais je crois que nous arriverons là en tout cas après le travail de la commission a un équilibre qui préserve celui souhaité par les différents auteurs de cette proposition de loi, je tiens à remercier, bien évidemment, les services de la commission des lois qui m'ont accompagné avec un rythme soutenu, au cours de ces quelques semaines pour pouvoir vous présenter le rapport et ce texte de commission ici ce soir et j'inviterais bien évidemment l'ensemble de mes collègues à voter favorablement. Et la parole est maintenant à monsieur Stanislas Guérini, ministre de la transformation et de la fonction publique. Monsieur le président, madame la présidente, ah ça, si ce le président Bazin, monsieur le président de la commission Jean Noël Buffet madame la rapporteure Cécile que mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, je veux le dire clairement et stratégique. S'agit de la capacité de la puissance publique à agir à répondre efficacement aux grands défis auxquels nous sommes confrontés et nous choisissons ensemble ce soir, c'est là nous nous rejoignons vous en remercier d'aborder ce sujet dans l'objectif de renforcer la puissance publique et sans jamais laisser ce sujet aux populistes. Je veux le dire les populistes ne cherche qu'une seule chose créé la polémique affaiblir le gouvernement se faisant, l'État et quand nous aurons proposer des solutions, ils passeront à la prochaine, ça n'est pas l'esprit des travaux que vous avez menée, ça n'est pas l'esprit du travail que nous mènerons ensemble ce soir, je souhaite que nous examinions ce texte dans l'esprit qui vous a animé de façon transpartisane, vous l'avez rappelé madame la précisant et présidente ou plutôt en étant rassemblés dans un seul camp, celui de ceux qui souhaitent renforcer l'État et sur ce sujet, la philosophie du gouvernement est claire est-ce que l'État doit pouvoir faire appel à des compétences dont tu ne dispose pas en interne, je crois que la réponse est oui, mais est-ce que l'État doit se renforcer, doit se réarmer doit développer ses compétences doit se doter d'un cadre renforcé pour recourir à des prestations ne concerne externe oui je réponds également positivement à ces questions là et je veux saluer en démarrant nos travaux, l'engagement du Sénat et de la commission d'enquête transpartisane créée à l'initiative, vous l'avez rappelé, madame la présidente du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste présidé par le sénateur Bazin et dont les travaux ont été rapportés par la présidente, ah ça, si vous avez mené un travail en profondeur précise sérieux avec des propositions concrètes sur le sujet, les membres de la commission ont estimé que ces propositions nécessité une traduction législative, le gouvernement en prend acte et nous travaillons sur ce texte de façon tout aussi attentive et exigeante et je me présente ce soir devant vous, avec la volonté d'avancer sur ces sujets. Et à l'appui de ses affirmations, je veux dire que nous avons agi concrètement pour encadrer le recours aux prestations de conseil, d'abord, vous l'avez rappelé avec la circulaire du Premier Ministre du 19 janvier 2022 elle a fixé, à la fois des modalités de contrôle interne et un cap en matière de réduction des dépenses de conseil à court terme, nous sommes en voie de tenir cet objectif, c'est aussi vrai des modalités de contrôle, je le dis devant la chambre haute, une mission inter inspection porté par la première ministre sera menée d'ici la fin de l'année pour vérifier la bonne application de ce point de contrôle interne et faire le point sur ce qu'il nous reste à faire, deuxièmement dès ma nomination, j'ai mis en place un nouveau cadre clair et renforcer sur le recours aux prestations de conseil c'est l'accord-cadre interministériel, porté par la DTP qui entrera en vigueur en janvier 2023 et sera d'utilisation exclusive pour les services de l'État, cet accord intègre pleinement les recommandations de la commission d'enquête en matière de déontologie en matière de transparence en matière d'encadrement des données ou de renforcement des risques contre les risques de dépendance des administrations vis-à-vis des prestataires, troisièmement afin de réarmer concrètement l'étage est aussi initier le renforcement de nos moyens humains, vous l'avez souligné madame la rapporteure en créant 15 postes dédiés au sein de la DTP pour une administration qui compte une centaine de fonctionnaires aujourd'hui, vous le verrez dans les engagements budgétaires dont vous aurez à débattre dans le cadre du projet de loi de finances, j'ajoute enfin un point très concrets, nous avons créé cette année, un document qui fait la synthèse de l'ensemble des dépenses de conseil de l'État et donc j'ai tenu bien entendu à ce qu'il vous soit rendue disponible avant l'examen de cette proposition de loi ce document annexé au PLF 2023 je prendre devant vous, 2 engagements concernant ce document d'abord c'est de porter un amendement dans le PLF 2023 dès l'examen du texte budgétaire à l'Assemblée nationale pour que ce document soit gravé dans le marbre et devienne un jaune budgétaire pour 2 bombes madame la rapporteure une annexe pérenne dans le cas de l'examen des des lois de finances que nous aurons à examiner chaque année le 2ème engagement, j'aurai l'occasion d'y revenir, dans nos débats c'est de renforcer le volume et la précision, la granularité des informations qui seront portés à connaissance dans ce jaune budgétaire, vous le voyez, nous avançons, nous agissons, nous prenons des expositions pour renforcer l'État en prenant en compte les recommandations du Sénat et c'est dans cet état d'esprit que je veux aborder la proposition de loi qui va occuper nos travaux ce soir dans un état d'esprit constructif sincère dans les finalités portées par ce texte et exigeant dans l'effectivité et la proportionnalité des dispositions que nous allons discuter ensemble, je vous le disais, je partage l'objectif 1er de ce texte meilleure maîtrise, par la puissance publique des moyens qu'elle mobilise et celui de neutralité des prestations de conseil sur la décision publique qui doit rester pleine et entière et je réaffirme tout l'intérêt de disposer d'un cadre légal clair et stable en la matière, un point de méthode pour nos discussions ce soir je vous dire les axes de travail que j'identifie pour renforcer le texte et je prends l'engagement pour les débats qui vont suivre, de toujours vous indiquer en transparence les points qui me semble soit inopérant soit disproportionnée et de toujours faire des propositions, je ne porte aucun amendement de suppression sentent contre-propositions, d'une certaine façon, que je souhaiterais vous soumettre les 3 sujets que j'identifie sont les suivants d'abord, vous l'avez mentionné Madame la rapporteure, le périmètre de la proposition de loi établie par l'article 1er j'ai beaucoup parlé de puissance publique je fait à dessein, car il nous semble essentiel de faire en sorte que le cadre proposé par l'article promener s'applique également aux collectivités territoriales, qui ont reçu aussi recours aux cabinets de conseil, nous aurons l'occasion d'en disputer d'en discuter et des amendements ont été portés en ce sens sur différents bancs dans cet hémicycle 2ème sujet sur la question de la transparence à la fois des prestations et des compétences de l'État, le gouvernement porte des amendements afin de recentrer en un article unique, les dispositions porté dans les articles 3 4 et 8, il s'agit de rendre, j'aurai l'occasion de vous présenter cette proposition plus claire, plus lisible et donc plus exploitable, les informations transmises par le gouvernement sur le recours aux prestations de conseil, enfin 3ème sujet sur le mécanisme de contrôle déontologique de sanctions, je souhaite que le contrôle exercé soit proportionnel à l'objectif poursuivi je crois très sincèrement que c'est une condition d'effectivité des mécanismes proposés nous aurons cette discussion pour les dispositifs qui concerne les déclarations d'intérêts exigés pour les consultants, mais aussi sur les mécanismes de contrôle de la HATVP et la question de la régulation des mouvements entre secteur public et secteur du conseil au fond, je viens de vous donner les 3 champs sur lequel j'aurais des propositions à formuler et sur lequel je souhaite surtout que nous ayons vraiment un vrai débat de fond pour nous assurer de la bonne effectivité de la loi, madame la présidente, vous m'interrogez au fond sur l'avenir de ce texte, j'ai la volonté que ce texte chemine, je l'ai dit publiquement, je le réaffirme ici devant vous sur les modalités de son examen, que ça soit dans le cadre d'une niche parlementaire, dont la programmation est à la main de chaque groupe ou sur le temps réservé au gouvernement, vous comprendrez qu'il est important pour le gouvernement que nous puissions examiner ce texte et de voir de quel texte on parle à l'issue des travaux que nous aurons ce soir, sur lequel la haute assemblée aura à se prononcer, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite que nous puissions maintenant rentrer dans le débat au fond, je crois que c'est ce que vous et moi attendons pour ce soir, je vous remercie. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Stéphane Ravier non-inscrits pour 3 minutes suivant l'usage. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues sur le ministre, vous êtes incorrigible la discussion générale n'a pas débuté que vous agitez déjà le chiffon rouge, véritable point Godwin du, il ne faut pas faire le jeu du populisme, ça traduit quand même une certaine fébrilité manque de sérénité du gouvernement mais que cela vous plaise ou pas, ce texte doit marquer la fin de très mauvaises habitudes pour l'état ou une collectivité territoriale, faire appel à un cabinet de conseil pour un soutien technique ou un état des lieux ponctuel, c'est légitime, y avoir recours de manière systématique et en devenir dépendants, c'est inacceptable, or, le Sénat a relevé un phénomène tentaculaire équivalent à une facture minimale de 1 milliard d'euros en 2021 pour l'État et ses opérateurs sont non seulement les proportions mais les méthodes qui interroge : nous comprenons désormais parfaitement ce que signifie la Start-Up nation. Un État colonisé par les cabinets, souvent étrangers comme les américains McKinsey ou Accenture ayant pour seul intérêt de faire de l'argent, bien loin des préoccupations d'intérêt général et encore moins d'intérêt national, la Start-Up nation c'est l'externalisation des missions régaliennes au profit des grands cabinets de conseil, la captation de notre souveraineté par le secteur privé et pas n'importe lequel, celui des plus fortunés des puissances étrangères et des grands lobbies financiers qui l'ont qu'une patrie, le profit, il est évidemment vital de mener une réflexion sur l'efficacité de nos administrations, l'effectif du ministère de la Santé s'élève à plus de 11000 personnes et il a fallu que le gouvernement mobilise plus de 11000 jours de consultant pour gérer la crise sanitaire, c'était insupportable cependant que nous n'ayons pas posséder en interne et les porte-flingue zélé de Los vaille sanitaire et vaccinal, ce n'est pas moi qui m'en plaindrait, ce sont les cabinets qui propose des solutions numériques de facilité, il parle en termes d'efficacité, pas de libertés de libertés publiques à trop les écouter les décisionnaires publics finissent par oublier les principes qui fondent notre état par ailleurs les cabinets conseils parfois simultanément plusieurs clients ils Servent les intérêts des plus offrant et renvoie l'ascenseur à ceux qui leur ouvrent les portes de Lino, de l'innovation de Pfizer a passé 25 ans chez McKinsey, cabinet chargé de la stratégie vaccinale en France cette porosité entre entre privés pose gravement problème parmi les ex-McKinsey en compte un préfet, le fils du président du Conseil constitutionnel, une vice-présidente de la région Île-de-France, un directeur de cabinet de ministre, le directeur général d'en marche et j'en passe 20 associés ont par ailleurs fait la campagne du candidat Macron en 2017, preuve d'une porosité public-privé politique très problématique, qui ne peut qu'entraîner défiance et suspicion avec le développement de structures comme le conseil de défense aujourd'hui, sanitaires, militaires et en attendant, environnemental et migratoires nous sommes sommés de prendre l'habitude dès huis clos, sans même un contrôle parlementaire ces manières d'agir de la part de l'exécutif ne doivent pas nous installer dans une forme d'accoutumance, il convient donc de rétablir les mécanismes de responsabilité et de légitimité propre, un système démocratique, il en va de la confiance des Français envers la politique qui est fortement éprouvée avec vous, mes chers collègues, je participerai à une avancée sans moi il dans ce sens. Et vous en remercie. Monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la rapporteure, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous avons tous en tête l'Estrie largement métallisé dès qu'ils auditions de la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés ou notre collègue rapporteur Éliane Assassi interroge l'un des dirigeants de McCain McKinsey France au sujet du un contrat d'un montant de presque d'un demi 1000000 d'euros, pour évaluer les évolutions du métier d'enseignant et la Direction interministérielle de la transformation publique dans ses réflexions autour du métier d'enseignant, un échange lunaire, tant du point de vue des montants évoqués que des réponses de celui qui était auditionné, alors je peux le dire sans détour toute critique que je pouvais faire sur ce texte ne sera cassé, soir et marginal au regard de la grande qualité et de l'intérêt supérieur des travaux qui ont été menées par notre assemblée sur un sujet essentiel, celui de la privatisation de la décision publique que par choix volontaire vers des cabinets de conseil, les travaux de la commission d'enquête nous ont placés face à 2 questions : celle de notre vision de l'État et de sa souveraineté face à des cabinets privés d'une part et la bonne utilisation des deniers publics, d'autre part alors de notre rate attachement profond à un État fort et garant de l'intérêt général, toutes les mesures de cette proposition de loi vont donc dans la bonne direction, qu'il s'agisse de la publication, en fait, de la liste des prestations de conseil auxquelles l'État et ses opérateurs font appel de l'encadrement plus contraignant du recours aux consultants ou encore du renforcement des règles déontologies des cabinets de conseil et des prérogatives de la haute transparence de la vie publique, bien sûr, un tel texte parce qu'il s'attaque à un sujet d'ampleur et complexe vient avec des difficultés, je pense en particulier à la détermination de ce qui doit être qualifié de prestations de conseil, l'article 1er de la proposition dresse une liste synthétique qu'il serait temps d'allonger par le détail des principes et des exceptions ce sens notre collègue Jean-Pierre Corbisez avait déposé un amendement en commission visant à exclure du régime du contrôle des prestations des entreprises d'ingénierie délivrées au titre d'une expertise technique cette précision n'était pas apparu superflu mais nous comprenons aussi qu'elle n'ait pas été retenu les auteurs de la proposition de loi et notre commission en fait le choix contraire de rester relativement souple dresser une liste exhaustive, leur a paru impossible nous ira joueront pour donner à ce texte, les chances d'une application rapide et finalement c'est le lot de toutes les qualifications juridiques que d'avoir des zones grises de laisser aux acteurs voir au juge le soin de les analyser de trancher au cas par cas, toutefois il irait à ce sujet qui pose une réelle difficulté ne nous plaisant à rappeler que notre assemblée représente les territoires, d'autant que la constitution par son article 24 nous en a donné la charge, vous savez déjà où aboutira mon propos, j'ai consulté quelques articles de presse sur l'examen de cette proposition de loi je n'incite cueille le Sénat oublie ses électeurs, la critique est évidente, mais surtout fondée en particulier à l'époque où la confiance, la décision politique autant à s'étioler je comprends évidemment les arguments qui ont conduit et sur les collectivités culotte local du périmètre de ce texte pour ne retenir que l'État et ses administrations, mais il donne le sentiment d'un refus d'obstacle notre président Jean-Claude Ruquier a déposé l'amendement qui permettrait de corriger cet écueil, il est curé de pour la première de cette proposition, les collectivités territoriales et la établissements publics, à l'exception des petites communes, ainsi que les intercommunalités, à l'exception des comités de communes, nous aurons le débat tout à l'heure, mais j'espère que nous ne nous cachons pas derrière les faux problèmes logistiques d'opérationnalité des seuils ou de mécanique juridique pour refuser cet aménagement nos collectivités elles aussi méritent d'être protégés de l'instruction excessive des cabinets de conseil des consultants dans l'élaboration de leurs politiques publiques chacun sait ici l'importance des décisions politiques prises sur nos territoires, le renforcement de la décentralisation a jusqu'à donner à nos collectivités pouvoir considérable entre pays, nous pouvons pas les exclure des réflexions sur la bonne utilisation des deniers publics, souvenons-nous du fameux précédent des emprunts toxiques dans beaucoup de collectivités ont été les victimes et qui un pays parfois encore le prix, les responsabilités étaient multiples, mais c'est aussi parce que des élus étaient mal protégés contre l'avidité de certains cabinets de conseil ou établissements bancaires qui n'ont pas pu prendre de bonnes décisions, toutefois je peux aussi le redire, le débat sur l'inclusion ou des collectivités n'enlève rien à l'intérêt et à la grande qualité du texte s'il faut l'adapter, que les collectivités soient incluses doctorant mais dans cette perspective, j'invite notre assemblée à poursuivre ses travaux, hein, s'engageant dans l'élaboration de régime un quadra également les collectivités. Merci, cher collègue, la parole est maintenant au président Arnaud Bazin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues comme Éliane Assassi je souhaite remercier tout d'abord, l'ensemble des membres de notre commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider, que de chemin parcouru depuis la réunion constitutive du 25 novembre 2021 il y a bientôt un an, notre rapport été transpartisan tout comme cette proposition de loi, c'est à la fois un gage de sérieux et d'équilibre partagé sur tous les bancs de l'hémicycle je salue également le travail de la commission des lois, qui a amélioré le texte et je remercie la rapporteure pour son écoute et sa connaissance du sujet que les choses soient claires, nous ne légiférons pas contre les cabinets de conseil dont nous ne remettons pas en cause le professionnalisme mais pour mieux encadrer leurs prestations et en finir avec l'opacité déplorée par la commission d'enquête, j'appelle aussi le gouvernement à inscrire notre proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, nos concitoyens ne comprendraient pas que ce texte se retrouve bloqué dans la navette parlementaire, cela ne serait pas à la hauteur des enjeux soulevés par la commission d'enquête, je vais concentrer mon intervention sur les aspects déontologiques, ce qui ne va pas vous surprendre. La commission d'enquête a mis en lumière 3 risques : les conflits d'intérêts, les cabinets de conseil conseil simultanément plusieurs clients dont les intérêts peuvent diverger la porosité lorsque les cabinets recrutent d'anciens responsables publics, ce que l'on appelle le pantouflage et enfin le pied dans la porte lorsque les consultants interviennent gratuitement pro Bono pour l'administration, ce sont par exemple les cabinet McKinsey, Boston Consulting Group qui ont organisé les sommets Tech for Good des choses France à l'Élysée, ces prestations était même devenu banal, alors qu'elle servait en réalité la stratégie commerciale des consultants avec cette proposition de loi, nous faisons, choix de la clarté, nous interdisons purement et simplement le pro Bono, ce que le gouvernement n'a jamais fait seuls resterait le mécénat. Dans les secteurs bien circonscrit comme l'humanitaire, la culture ou l'éducation, pour plus de transparence, le mécénat, ferait l'objet d'une déclaration à la Haute autorité pour la transparence, tout comme les actions de démarchage ou de prospection commerciale des cabinets de conseil dans la même logique, nous souhaitons que le cabinet de conseil, et les consultants remplissent des déclarations d'intérêts sous le contrôle de la Haute autorité, l'État est en droit de connaître les autres clients de ces consultants afin de mieux prévenir les conflits d'intérêt et surtout d'y mettre fin, un État aveugle sur le plan déontologique est un État en danger, l'enjeu n'est pas mince au regard des récentes interventions des consultants sur la crise sanitaire, ou encore l'évaluation de la stratégie nationale de santé. Des consultants ont fait part de leurs inquiétudes dans la presse, les déclarations d'intérêts seraient trop lourdes et les forcerait à s'éloigner du secteur public, qu'ils se rassurent, il se rassure en tant que parlementaires, nous remplissons des déclarations d'intérêt depuis 2013 la première prend un peu de temps, puis il suffit de l'actualiser, je pense que des bac plus dix y parviendront sans grande difficulté. Tout ça est loin d'être insurmontable, je pense que les collègues ainsi que vous Monsieur le Ministre, vous pourrez le confirmer, il en est de même pour le pantouflage, nous n'empêchons pas les consultants d'aller travailler pour l'administration, et réciproquement, en revanche, nous souhaitons que l'avis de la Haute autorité soit systématique et que l'intéressé lui rende compte de son activité à intervalles réguliers pour vérifier que les exigences de la Haute autorité sont bel et bien respecté, rien d'insurmontable encore cela évitera par exemple qu'un consultant de Cap Gémini soit embauché au service des correspondances de l'Élysée et recrute ce même cabinet pour moderniser le service toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est bien sûr pas fortuite. Dans un souci d'efficacité, nous souhaitons renforcer les moyens d'investigation et de sanction de la Haute autorité, cette dernière doit pouvoir prononcer des sanctions administratives en cas de manquements déontologiques des consultants, ce qui évitera d'engorger les tribunaux, elle pourra aussi les exclure de la commande publique, ce qui nous semble logique et conforme au droit européen, vous voyez mes chers collègues, que nous proposons un dispositif déontologique à la fois complet et cohérent, mettant en oeuvre les recommandations de la commission d'enquête ou que vous viendrez que la confiance de l'administration envers ces consultants n'exclut pas le contrôle, ce qui justifie notre proposition de loi je finirai en évoquant les représentants d'intérêts, ce sujet n'entre pas dans le périmètre notre texte, comme l'a justement rappelé la commission des lois. Je n'ignore toutefois pas son importance ni la nécessité de faire évoluer le droit en vigueur, c'est dans cet esprit que le comité de déontologie du Sénat présentera des propositions sur les représentants d'intérêts d'ici à la fin de cette année, après avoir entendu les professionnels du secteur, nous l'avons commencé depuis bientôt un an et les associations, c'est un engagement que nous avons pris auprès du bureau du Sénat et que nous tiendrons je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien à notre proposition de loi. Et la parole est maintenant à Emmanuel Capus pour le groupe, les indépendants.

Monsieur le président, sur le ministre. Mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi issu des travaux de la commission d'enquête menée à l'initiative de Madame la Présidente, assassiné. Cette commission d'enquête trouve son origine dans une polémique née à l'occasion d'élections présidentielle présidentielle. Polémique concernant le recours du gouvernement au cabinet de conseil. Certains de nos concitoyens ont en effet été interpellé par le fait que l'État, recours à des cabinets privés pour l'aider à définir sa stratégie. Mes chers collègues. Cela a été dit d'ailleurs par le président Bazin aussi divers que soient ses services, l'administration n'a pas et ne peut pas avoir en interne les compétences requises pour faire face aux situations qu'elle doit gérer. Le recours à ces cabinets permet donc d'apporter une expertise et de proposer des solutions. C'est ainsi que 72 % des prêts des 900 millions d'euros dépensés par l'État en conseil durant l'année 2021. Concerne des prestations informatiques. Tous les responsables politiques savent bien qu'ils ont eu recours aux prestations de conseil. Ou qu'il y auront recours un jour. Et nos concitoyens français préfèrent sans doute que l'État prenne des décisions éclairées. La proposition de loi que nous examinons vise à imposer des obligations de transparence aux prestataires de conseil lorsqu'il travaille au bénéfice de l'État et de ces établissements. Afin de prévenir les conflits d'intérêt mais aussi afin d'éviter les allers-retours entre ces cabinets et l'administration. Pour cela, le texte étant le pouvoir de la Haute autorité pour la transparence de la vie politique, déjà en charge du contrôle des principaux responsables et agents publics ainsi que des lobbies. L'état. N'est évidemment pas le seul à recourir aux prestations de conseil nos régions, nos départements et nos communes le font aussi très régulièrement. Pour des raisons de périmètre d'enquête, cette proposition de loi ne vise cependant pas les collectivités territoriales. Certains parmi nous s'interroge cependant sur la nécessité d'inclure les plus importants d'entre elles dans ce dispositif. En vérité, notre groupe s'interroge plus largement sur l'opportunité d'une telle loi. Nous comprenons parfaitement les inquiétudes que l'activité de conseil a pu susciter mais nous doutons que les moyens proposés soient efficaces et adaptées. L'administration fait appel à de nombreux acteurs afin d'avoir un oeil extérieur pour résoudre les difficultés auxquelles elle est confrontée. Nous croyons, mais manifestement nous sommes minoritaires et qu'il n'est pas malsain que publiques et privées puissent échanger des idées et des personnes. Par ailleurs, quels que soient les conseils. C'est toujours mes chers collègues, le responsable politique qui décide. Et qui est responsable des décisions qu'il prend. Cela vaut également pour celle de recourir au Conseil. Nous ne sommes donc pas favorable à la création de régimes spécifiques dont l'application est confiée à des autres. Autorité spécifique qui disposerait de pouvoirs d'enquête et de sanction spécifique. Enfin, nous craignons que cette PPL ne renforce des mots très français.

ça peut intéresser certains évidemment. Nous sommes convaincus que notre pays a au contraire besoin de souplesse et de simplicité, les échanges public-privé, sont monnaie courante dans beaucoup de pays et dans ceux du nord de l'Europe, particulièrement. Il ne s'en sort pas plus mal, c'est fertilisation croisée sont créatrices de synergies qui améliore l'efficacité de l'action publique. Bien sûr, nous devons être très attentif aux ressources de l'administration, elles proviennent de l'argent des Français et doivent donc être employé à bon escient. Et sans abus, cela va sans dire. Mais nous croyons qu'il faut également veiller à préserver son efficacité. Si nous ne voulons pas travailler nous-mêmes à l'impuissance de l'administration. Le gouvernement a annoncé son intention d'encadrer davantage le recours aux prestations de conseil par les administrations publiques, et c'est une bonne chose. Pour voir. L'une des manières de réduire ce recours, la plus efficace. Pour les libéraux que nous sommes. C'est certainement de réduire le périmètre d'action de l'État, qui pourra ainsi se concentrer sur ses missions régaliennes. Ses missions les plus essentielles et sur lesquels il dispose d'une vraie expertise. Dans sa majorité, vous l'aurez compris le groupe les en défendant ne votera pas comme Monsieur Ravier ni comme certains autres sur ce bon et s'abstiendra. La parole est maintenant à Guy Bénard roche pour le groupe Écologie Solidarité territoire. Et pour cinq minutes.

la fin du pantouflage des allers-retours trop opaque entre les hautes sphères de l'État et les cabinets privés avaient été clairement érigée en objectif par notre président, Emmanuel Macron. Comme cela devient une habitude des gouvernements, du président de la République. En quelque peu déçu sur ce programme, malgré l'espoir de nos concitoyens sur la réelle prise en 2 ans Côte du devoir d'exemplarité mais comme pour d'autres décisions de cette gouvernance, je cite : ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché. C'est ce que dit couramment notre président de la République, c'est lui-même qui l'a dit, pour d'autres. La présente proposition de loi s'inscrit dans l'histoire récente des révélations journalistiques d'une augmentation notable des dépenses liées au cabinet de conseil depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, le groupe CRCE avait alors demandé l'ouverture d'une. Enquête sur l'affluence de ces cabinets et la présente proposition de loi s'appuie, Monsieur le Ministre, sur les conclusions de cette commission transpartisane, rendu au printemps 2022. Quels sont les reproches formulés à cette explosion des recours quoi c'est privé mais surtout quelles sont les propositions que porte cette loi pour y faire face. Tout d'abord ce n'est pas le recours même à une. Extérieure qui est mis en cause mais bien les mécanismes qui amène la transparence nécessaire à ces contrats et les montants consacrés pour parfois des résultats plus que discutable le désinvestissement dans la fonction publique qui ne résulte pas seulement de l'action de ce président, il faut l'avouer, mais aussi de ses prédécesseurs, contribue à ce recours massif, les sociétés de conseil sont souvent perçus comme un moyen simple et Agile dans les moments de surcharge ponctuelle pour palier au plafond d'emplois cela crée en conséquence des pertes de compétences ou c'est de l'administration ou quelques fois l'empêchement de la montée en compétence l'exemple typique : on est la compétence informatique. Certains y voient d'ailleurs l'action de pompier pyromane qui ne donne pas les moyens à l'administration de rester compétente sur ses prérogatives dans le but de justifier ces recours coûteux à une poignée de grosses entreprises de conseil. Pourtant, une grande majorité des entreprises de conseil de moindre échelle reste loin du pouvoir et des pratiques de ces grands groupes. Cette dynamique de recours des. Couplée au cabinet de conseil est aussi critiqué dans son manque de transparence, résultats d'études coûteuses Éliane Assassi nous l'a rappelé non publiés, par exemple dans l'Éducation nationale. Doublant de mission, vous l'avez également rappelé, privé, public, par exemple pour la prise en charge de la petite enfance. Cette opacité dans le recours, que ce soit dans la définition du besoin réel ou dans l'effectivité réelle des rendu et source de défiance de nos concitoyens, y compris dans notre système démocratique. Au vu de toutes les problématiques, révélées par la commission d'enquête sénatoriale qui, au delà de marquer les dérives a pu proposer 19 recommandations notre collègue a donc souhaité travailler la proposition de loi que nous vous proposons aujourd'hui. Si nous apprécions ce texte. Nous pensons que certains points méritent, si ce n'est amélioration au moins une discussion. Je tiens par exemple, au nom de mon groupe, a regretté la décision d'recevabilité qu'ont subi nos amendements, alors qu'ils concernaient explicitement les pouvoirs de contrôle et de sanction conféré à l'autre autorité pour la transparence de la vie publique en vue de faire respecter ses obligations par les prestataires de conseils, les consultants, comme indiqué dans le document de la commission des lois, qui fixe les règles relatives à l'application de l'article 45 un de ces amendements est recevable s'inscrivait de plus dans la lignée d'une recommandation de la mission d'évaluation de la loi sapin de mener en 2021 par 2 députés, Olivier Martin des républicains et Raphaël Gauvain de la République en marche dans sa proposition numéro 42 du rapport d'évaluation, il ne faisait en plus que répondre à une demande même de la HATVP qui est explicitement dans un rapport d'octobre 2021 à sa proposition numéro 12 demander de doter la Haute autorité de pouvoirs propres de sanctions administratives en cas de manquement à l'obligation de dépôt d'une déclaration d'activité, la sanction étant proportionnée à la gravité du manquement et à la situation de la personne poursuivie, nous le regrettons vivement déjà ce périmètre nous apparaissait particulièrement resterait ne permettant pas une discussion globale sur les lobbies et les Liad atterré entre public et privé, notre groupe est certes minoritaire et dans l'position hélas parfois aussi, mais le refus la discussion au travers de décision irrévocable d'irrecevabilité pénalise. L'exercice démocratique et le l'autre pour en revenir au texte, ces mesures novatrices douze ils sortent globalement favorable. Pour autant, la plupart des dispositions de sa PPA, elle s'endort normative, mais certaines d'entre elles revêtent un caractère réglementaire, elles ont donc pour objectif d'inciter le gouvernement à opérer des changements dans les règles déontologiques, c'est bien là que le bât blesse, tout comme dans l'lors de la création de la HATVP, c'est l'écriture des décrets qui, parfois, de suite, c'est pourquoi nous aurons à coeur de discuter et d'entendre les gages que donnera le gouvernement pour de réelle transformation de ce recours excessif au cabinet de conseil les gages pour permettre à la HATVP de pouvoir fonctionner correctement et notre groupe votera pour ce projet. Merci, cher collègue, et la parole est à Nicole Duranton pour le groupe RDPI. Et pour ces minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, chers collègues, les pouvoirs publics ont toujours eu besoin de s'appuyer sur des compétences extérieures, c'est une réalité ancienne qui ne date pas uniquement depuis l'élection présidentielle de 2017 mais déjà depuis de nombreux quinquennat et s'est accélérée depuis 2007 RH, informatique, gestion de données massives communication analyse comparative, les besoins sont en réalité nombreux pourquoi d'abord certains champs d'expertise très très spécialisés, le nécessitent ensuite un arbitrage apaisé appelle parfois un regard extérieur, enfin l'urgence ou le lancement d'un projet implique l'action rapide et coordonnée d'un grand nombre de consultants agissant uniquement dans un laps de temps déterminé ce qui se prête mal au processus de recrutement de fonctionnaires pour autant le besoin ne sera pas toujours aussi important que durant la crise Covid d'une part, nous avons vécu ces dernières années dans une accumulation de crises globales tout à fait inédite, d'autre part, chaque administration travaille son attractivité afin de recruter en interne ses compétences, je voulais également souligner que nous ne nous ne sommes pas les plus mauvais élèves en Europe, ainsi en 2018 : un rapport souligne que, comparé aux autres pays européens, le conseil au secteur public apparaît limité en France, les chiffres sont 5 fois plus élevé en Allemagne et 4 fois plus au Royaume-Uni la résolution numéro 111 a été enregistrée à la présidence du Sénat le 27 octobre 2021, une commission d'enquête a ensuite été constituée donc cette commission dont j'étais membre entendu pendant quatre mois 47 personnes sous serment lu les réponses à 131 questionnaire et analysé 7300 document comme mes collègues l'ont déjà, souligne le rapport a été rendu le 16 mars dernier et je salue le fait que le gouvernement est pris en considération les recommandations lors de les lobes à l'élaboration du nouvel accord cadre plafonnant les dépenses de conseil renforçant la transparence et améliorant l'évaluation par ailleurs, le gouvernement a d'ores et déjà publié un jaune budgétaire annexé au PLF 2023 et intitulé recours au Conseil extérieurs, il s'agit là d'un pas supplémentaire vers plus de transparence compétents souveraineté démocratie et légitimité de la décision voici autant d'enjeux que cette pratique implique et qu'il convient de sécuriser le 1er ministre avait déjà publié le 19 janvier une circulaire portant l'objectif ambitieux de diminuer de 15 % le volume de prestations de conseil en stratégie, en 2022 toutefois les dispositions concernant la transparence mérité d'entrer dans le Champ législatif, je salue le travail préalable en 2014 et 2015 des rapporteurs pour information de la commission des finances sur la communication de la Cour des comptes, le mercredi 12 octobre la commission des lois, adoptées à l'unanimité la PPL, cabinet de conseil tous les amendements de la rapporteure ont été adoptées également cette proposition de loi vise à traduire dans la loi les préconisations de la commission d'enquête, assurer la traçabilité de la participation des cabinets et garantir une meilleure information des citoyens, mais en aucun cas à supprimer le conseil notre groupe le RDPI souhaite apporter quelques modifications au texte en déposant 5 amendements, le premier amendement que nous proposons, précise dans l'article 1er le seuil des établissements publics concernant par le chant de la PPL, en effet, il est essentiel d'éviter de faire peser une charge déraisonnable sur des structures de taille réduite, 60 millions cela correspond au seuil des avances obligatoire versée aux PME dans le cadre d'un marché public, seuil déjà bien connu des acteurs concernés, le second vise à exclure les prestations des conseils, un terme à l'administration pour éviter une sur-interprétation par le juge le 3ème réaffirme l'exclusion des prestations de gestion RH et d'expertise informatique concernant l'article 11 nous portons un amendement pour que les modalités d'enregistrement des actions de démarchage soit défini par décret, l'objectif étant d'aligner le dispositif sur les règles de droit commun, enfin sur l'article 18, il s'agit de limiter les obligations d'audit souvent très coûteuses au marché les plus sensibles qui le nécessitent, durant les travaux de la commission a été développé l'idée d'appliquer le dispositif aux communes, collectivités territoriales, en effet, les régions, les départements, les EPCI et certaines villes font aussi appel au Conseil et cela s'inscrit dans la suite logique des choses, toutefois, cette extension du Champ de la loi doit passer par la fixation d'un seuil, le gouvernement et plusieurs collègues des différents groupes ont déposé des amendements portant ce seuil à 100000 habitants se chiffrent semble tout à fait adapté, je sais que notre Ministre Stanislas Guérini aura à coeur de ne pas dévitaliser le texte de la commission, il convient de rendre visible l'action de chaque acteur des politiques publiques, d'empêcher toute dérive mais aussi de ne pas tomber dans la surenchère législative de ne pas ajouter aux différents niveaux, une surcharge de travail et des règles règles confuses, le groupe RDPI est favorable sur le principe de cette proposition de loi, nous serons très attentifs au vote des différents amendements, le texte issu des travaux de la commission est équilibré et s'inscrit dans la continuité logique des travaux de la commission d'enquête, il sera nécessaire de veiller à ce que le dispositif puisse facilement être mis en place par l'administration, on l'alignant le plus possible sur ce qui existe déjà pour les représentants d'intérêts, je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mais monsieur le Président Madame la rapporteure, chers collègues, je voudrais d'abord au nom du groupe socialiste remercier très sincèrement nos collègues Éliane Assassi et Arnaud Bazin. Pour avoir fait avec tous les membres de la commission d'enquête, un travail tout à fait remarquables et ce travail remarquable illustrent une fois encore, mes chers collègues, combien le Parlement et particulièrement le Sénat peut être utile et efficace lorsqu'il exerce pleinement la mission de contrôle qui lui est dévolu par la Constitution, donc merci pour ce travail, ce travail a permis notamment l'ouverture d'une enquête judiciaire suite à la découverte du non-paiement d'impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020 par le cabinet McKinsey, alors qu'il réalise en France un chiffre d'affaires annuel de plusieurs centaines de millions d'euros, c'est inacceptable. Impossible que cela continue ainsi, nous avons également grâce à la commission d'enquête découvert que l'État avait dépensé en 2021 plus d'un milliard d'euros on peut prestations de conseil de cabinet privé 45 pour qu'en 2018 nous avons découvert que par rapport à la crise sanitaire, il avait été fait largement conseil appel à ces cabinets or mes chers collègues, nos services, les services de l'État dispose de compétences considérables. Et il est parfois regrettable que l'on fasse appel à des instances priver alors que les services publics disposent des compétences nécessaires, je voulais dire aussi que, un jour. J'ai appris. Qu'un ministre avait fait appel à un cabinet de conseils pour rédiger l'exposé des motifs d'une proposition de loi d'un projet de loi, c'est absolument insupportable si un ministre ne peut pas rédiger les raisons pour lesquelles ils présentent. Une un projet de loi, alors c'est à désespérer de la politique, donc ne mélangeons. Pas tous, il est vrai qu'il est des domaines dans lesquels il est utile de faire appel à des compétences extérieures à l'administration, personne ne le conteste, mais encore faut-il que ce loi ce que cela soit fait en toute transparence, alors mes chers collègues, nous avons déposé nous aussi quelques amendements pour élargir le Champ, alors je sais bien qu'on nous a dit Madame la rapporteure, vous nous avez dit : finalement, il nous est apparu plus sage de nous en tenir strictement au Champ de la commission d'enquête, j'entends cet argument, mais rien n'empêche le législateur que nous sommes, d'aller plus loin, absolument rien, et si les principes sont bons. Au terme des travaux de la commission d'enquête pourquoi. Ne pas élargir le Champ, c'est pourquoi nous avons nous aussi penser aux collectivités locales d'une certaine importance, chers collègues, plus de 100000 habitants, nous avons pensé à la Caisse des dépôts et consignations et nous avons aussi pensé aux assemblées parlementaires parce qu'enfin, ne serait-il pas logique que nous appliquions à nous-mêmes les excellentes, règles qui ont été formulées dans le rapport, c'est une question alors nous savons déposé un amendement en prenant soin dans sa rédaction, j'insiste là-dessus qu'il préserve intégralement l'autonomie des assemblées parlementaires, c'est-à-dire que c'est le bureau de chaque assemblée qui décidera des modalités de mise en oeuvre, en tout cas, il nous ça paraît, on pourra en discuter bien entendu et diverses méthodes sont peut être possible pour atteindre ce but, le but c'est quoi, c'est la transparence et nous avons grand intérêt dans ce domaine, comme beaucoup d'autres, a joué la carte de la totale transparence à l'égard de nos concitoyens, il est un livre très ancien qui a connu quelques succès et je terminerai là-dessus monsieur le président, et Madame la rapporteure, dans laquelle on peut lire cette phrase : la vérité vous rendra libre, je vous remercie. Merci et là. Parole est à monsieur Éric Bocquet pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour également cinq minutes. C'est le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les cabinets de conseil privés, acteurs de l'ombre omniprésent pourtant tentaculaire, a jugé la commission d'enquête sénatoriale ont été démasqués dévoilés mis au grand jour les parlementaires du groupe CRCE sont à l'origine, ils ont conduit par le biais de notre président, avec les membres de la commission d'enquête, et le président Arnaud Bazin une investigation qui, je le dis nous a dépassé nous a dépassé d'abord par la résonance populaire que les travaux ont eu les cabinets de conseil constitue désormais un objet politique identifié et controversée, nous devons collectivement nous en féliciter. Elle nous a dépassés aussi par l'impérieuse nécessité de légiférer rapidement, c'est ce que nous faisons ce soir pour traduire en actes les constats partagés par les membres de la commission d'enquête à l'unanimité. Si le recours à des cabinets de conseil est ancien, son ampleur est inédite : un milliard d'euros en 2021 ce qui diffère d'hier, c'est surtout une croyance toujours plus affirmée qui transparaît depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas les sachant étant les cabinets de conseil et les autres sont dans l'administration. Le monopole de la vérité objective et rationnelle incomberait à des cabinets connu pour appliquer à des problèmes différents les mêmes recettes : économies d'échelle oblige. Nous nous souvenons des mots de Nicolas Sarkozy, ancien prudent de la République le 12 décembre 2007, dès les premiers mots de sa présentation de la fameuse révision générale des politiques publiques, je cite : la réforme de l'État, je l'ai promise, je la ferai, je la ferai parce que nos finances publiques doivent être redressé ces mots matérialisée par le nom Laurent non remplacement d'un fonctionnaire sur 2, ont porté un coup important à la capacité de la fonction publique, de mener à bien ses missions. Chacun reconnaît aujourd'hui que la dérive est allé beaucoup trop loin, il faut consacrer le retour du politique comme maître de l'action publique, nous fûmes bien les seuls à proposer dans le cadre de l'examen de la révision de la LOLF le du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, la suppression de la fongibilité asymétriques terme barbare qui permet de redéployer le budget du personnel vers des dépenses différentes investissement intervention ou Consulting, entre guillemets, permettez-moi cet anglicisme, mais qui interdit le mouvement inverse cette logique libérale et mortifère, je souhaite que tous nos concitoyens et nos concitoyennes défi ces mécanismes libéraux de réduction de l'emploi public, au prétexte de prétendues obésité de l'État, le collectif nos services publics, explique cet effet pervers de diminuer le coût du service tout en maintenant sa qualité on en réduit la qualité tout en dégradant les finances publiques, fin de citation par le fait, notamment, de rémunérations beaucoup plus élevées pour les cabinets de conseil. Feignant de soutenir la proposition de loi transpartisane du Sénat le gouvernement et ses alliés révèlent leur volonté de miner le texte quelque part à grands coups d'exclusion et de suppression, on ne peut pas prétendre encadrer le recours aux cabinets de conseil en même temps leur faire béatement confiance, on ne peut pas prétendre encadrer les cabinets de conseil et en même temps, exclure des consultants au titre de leur statut, on ne peut pas prétendre encadrer le recours aux cabinets de conseil et en même temps, saper les obligations déontologiques que prévoit la présente proposition de loi des pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, mais votre en même temps on n'est pas l'équilibre c'est le laxisme, c'est la poursuite de la connivence entre le cabinet de conseil et le gouvernement des contrats massifs passé durant l'été et en ce début d'Automne monte que vous n'avez tiré jusqu'ici aucune leçon sur le fond des travaux de la commission et entendez bien vous limité à des déclarations d'intention tout au long du processus, vous n'avez eu de cesse de miner les travaux de la haute assemblée, sentant tant que la situation vous échapper quelque peu publication d'un rapport à l'Assemblée circulaire opportune la veille d'une audition du ministre, conférence de presse de ministre en pleine campagne présidentielle et publication d'un jaune budgétaire incomplet avant même le vote de la proposition de loi les mots du président, alors candidat sont teintés de vérité sur McKinsey on est mauvais comme des cochons, les enfants, je prends un instant car vous connaissez mon appétence en matière de lutte contre la fraude fiscale et toutes les formes d'optimisation intolérable, la commission a prouvé que McKinsey ne payait pas d'impôt sur les sociétés depuis 10 ans, alors même que celle qu'on appelle la firme réalisé plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année et capté de l'argent public merveilleux Weir, qui compte 970000 habitants et un 1000000 600 1000 sociétés enregistrées, chers collègues, nous sommes fiers de ce texte, fier de l'esprit de construction transpartisane qui nous a animés, c'est un point de départ bienvenue pour celles et ceux qui pensent encore que l'État peut et que l'État doit garantir l'intérêt général. La parole est à présent. Ah madame Nathalie Goulet pour l'Union centriste. J'ai pris des Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, arrivé en 9ème position, beaucoup de choses ont déjà été dites, je voudrais revenir sur sur nos travaux avec quand même une petite aigreur c'est de pas avoir eu l'idée moi-même de cette commission d'enquête, j'en ai une très grande frustration et je remercie Éliane Assassi et son groupe d'abord eu cette idée que je n'avais pas eu, je m'étais limitée lors d'un rappel au règlement à un débat sur le sujet, et voilà que la commission d'enquête est arrivé le sujet mérite et les travaux de notre commission d'enquête dont j'ai eu l'honneur d'être vice-président sont le le témoin mérite qu'on s'y soient penchées, le sujet est important au au plan financier, la part du privé dans la décision publique, dans quelles conditions sous quelles garanties, c'était un sujet qui n'est pas que philosophique dans notre société est friande, est ouverte au au conflit d'intérêts qui sont à mon sens le pire, cancer de la politique, encore une fois, il n'a jamais été question d'interdire le recours au cabinet conseil mais 2 encadrer ces recours pour plus de transparence afin d'assurer une plus Value réelle sans l'interdire, on peut s'interroger sur le fait que l'état de plus en plus recours à ces cabinets, y compris pour les politiques publiques les plus sensibles, c'est une tendance à à ubérisés le pouvoir régalien qui est de mon point de vue relativement inquiétante, c'est une philosophie dont certains dont je fais partie, on difficulté à à accepter placardisé la haute fonction publique en lui préférant à prix d'or des cabinets extérieurs privés c'est dévaloriser s'est paupérisé la haute fonction publique et les inspections générales, dont nous savons très bien qu'elle regorge de compétences souvent et rarement écoutés ou entendus en page 39 du rap en page 39 du rapport, vous avez une déclaration de Martin Hirsch, qui a confirmé le malaise que peuvent ressentir les agents autant le fait de travailler, y compris dans le corps médical sur un projet donné avec un regard extérieur ne pose aucun problème, autant le fait d'avoir une sorte d'abonnement auprès de grands cabinets de consultants et de personnes pour lesquelles l'hôpital n'est qu'un client. N'était pas perçu Pauline positivement en page 13 du rapport, les agents de l'Ofpra, déclare ainsi : j'ai l'impression que nous sommes régulièrement infantiliser, il faut rappeler qu'un cabinet conseil pour ce sujet et fournissant une prestation pour réduire les délais de traitement des demandeurs d'asile, délai qui n'est toujours pas réglé d'ailleurs aperçu à 485818 euros, la valeur ajoutée n'est pas immédiatement perceptible moderniser ce n'est pas paupériser paupériser comme moderniser notre diplomatie n'aurait pas dû être un petit matin d'un petit lundi de Pâques, de supprimer la fonction de le corps diplomatique, ni de supprimer l'ENA, dit le corps préfectoral, au 1er janvier 2023 je ne crois pas à ces réformes en faut qui ne sont que des réformes en trompe l'oeil d'ailleurs jamais évaluer donc le sujet n'est pas uniquement technique, il est politique et donc c'est à juste titre, locaux, le groupe CRCE pencher le gouvernement a d'ailleurs été contraint de réagir face aux travaux menés en toute transparence avec des auditions, ouvertes au public, ils sont toujours en ligne le 19 janvier 2022 sous la rubrique il faut sauver le soldat Montchalin, une circulaire a été publiée le matin même de l'audition, même pas la veille pour limiter le recours des ministères au cabinet conseil circulaire insuffisante mais attestant. De la Jeanne, on peut se le dire, on est entre nous, il est tard du gouvernement face aux effets de nos auditions publiques, bon, un mot sur le périmètre, alors là je suis prise une double sincérité franchement centriste, il est évident que la la question des collectivités locales se pose se pose, il y a pas, il y a pas de volonté de ne pas traiter la question des volontés de des des collectivités locales, mais pour les régions, les départements, les grandes métropoles, les intercommunalités, c'est un sujet. à part entière et nous ne l'avons pas traité durant notre commission d'enquête, nous n'avons pas eu une seule audition sur le sujet, nous n'avons consulté aucune des associations d'élus, c'est pourquoi notre groupe sur ce sujet, ça peut s'abstiendra sur les amendements pour une raison très simple, hein, ça n'a pas été traité lors de la commission d'enquête, mais surtout les associations d'élus n'ont pas été consultés, et donc de notre point de vue, il est tout à fait inacceptable de les, de les intégrer dans ce dispositif, sans avoir été entendu notre commission d'enquête a clairement défini le périmètre la loi encadre enfin la proposition de loi est cadré sur les travaux de notre commission d'enquête, les collectivités locales, je vous l'accorde, monsieur le ministre et j'accorde à mes collègues qui ont déposé les amendements, c'est un vrai sujet, je pense que de ce point de vue là on pourra avoir une autre mission, une mission flash Monsieur le Ministre, vous pouvez nommer quelques parlementaires en mission sur le sujet, on pourra d'ailleurs travailler aussi sur les centrales d'achat, ce sera aussi important sur les prestations de conseil et le recours aux cabinets d'avocats, le Conseil national des barreaux s'est vanté sur les réseaux d'avoir obtenu un résultat et d'être exclue du périmètre de contrôle, voilà le le tweet mortifère nous du du Conseil national des barreaux, nous venons de faire modifier la proposition de loi sur l'encadrement des cabinets dit de conseils cette proposition sénatoriale, prévoyez d'englober dans son périmètre, les prestations de conseil juridique, oui, mais enfin Monsieur le Ministre, vous savez que sur les directives européennes, nous avons eu exactement le même type d'irritants lorsque des cabinets d'avocats monte. Sujet cher à à mes collègues du groupe communiste républicain et citoyen et à Éric Bocquet, tout un tas de pyramide pour faire de de l'optimisation, voire de les de de la fraude fiscale, il était évident qu'il fallait les rentrées dans les dispositifs légaux, donc bon le texte et comme ça, pour l'instant, mais je pense que sur ce sujet, il faut travailler faut sera faut travailler avec les bâtonniers il faut travailler dans le domaine réglementaire, et il faut améliorer les dispositifs de transparence, vous ne pouvez pas consulté un cabinet d'avocats sur la loi sur les mobilités en ignorant absolument s'ils sont ou pas, l'avocat de telle compagnie de Vélib ou de telle autre société pour lequel il y aurait, sinon des conflits d'intérêts, du moins des Liens d'intérêts qui posera un certain nombre de problèmes, je pense que ce sujet est un sujet extrêmement important et et qu'il faut le traiter parce que, encore une fois, comme j'ai dit au début de mon intervention, le conflit d'intérêt et de mon point de vue là le le pire, cancer de la vie publique, alors un petit mot sur l'article 8 quand même qui va provoquer quelques remue-ménage c'est des nouveaux évidemment pouvoir de la Haute autorité de la transparence de la vie publique, bon moi je considère que c'est une bonne disposition

ni avec le Commissariat au Plan. Et je dois dire que ce défaut d'articulations nous a laissé un tantinet songeur donc le rapport fourmille de 7300 document 4 millions d'euros pour McKinsey 41 millions pour 68 commandes pour la crise sanitaire 485000 euros pour l'étude sur la réduction du temps des attentes des demandes d'asile dont on sait très bien que ça n'a pas du tout fonctionné sans parler de McKinsey, agent de liaison entre l'État et les agences de santé publique pour 169440 euros pour cinq mois d'études, tout cela, nous ne sommes pas du tout, raisonnables, je pense que cette commission d'enquête est une excellente plus-value pour notre haute assemblée que c'était, c'est une autre plus-Value pour le travail parlementaire et c'est une autre plus-Value pour le travail républicain que nous menons, je vous remercie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le président de la commission d'enquête, madame la rapporteure du texte et même le rapporteur de la commission d'enquête, mes chers collègues pour reprendre Talleyrand suffisant. Est insuffisant, c'était un l'attitude du gouvernement lorsque cette commission d'enquête a été créée, elle les lorsqu'elle a rendu ses conclusions. à l'époque, votre prédécesseur, monsieur le Ministre. Ah, fait fi un peu de nos remarques, j'ai même entendu à l'époque un jeune et sémillant porte-parole du gouvernement que de toute façon cette enquête avait été faite par une rapporteur communiste je, je, je l'entends encore à la radio le dire, oubliant par là même que ce rapport avait été adopté à l'unanimité du Sénat et donc ici avec des collègues de tous les bancs, bon c'est pas grave, c'était une erreur de plus et cette erreur, elle n'a, il n'a pas été de tenter de la corriger, effectivement, cela a été rappelé par mes collègues précédemment qui une circulaire le jour ont commencé à la commission d'enquête qui un autre rapport ailleurs qui le jaune maintenant, bon, on voit bien que on court un peu après tout ça, on n'est pas très à l'aise, hé bien, nous rassurez-vous. On n'est pas là pour accuser les uns ou les autres, on est là pour faire notre travail de parlementaire en lien avec l'exécutif, en lien avec l'administration qui va donc devoir se priver un petit peu de ces cabinets de conseil alors rassurez-vous, le Sénat est absolument pas contre l'utilisation des cabinets de conseil, notamment en matière informatique, voilà des choses que l'on apprend on en en faisant beaucoup alors quand vous menez un seul projet informatique important dans une administration, hé bien vous n'avez pas cet apprentissage, mais ce n'est pas le cas, mes chers collègues de la haute fonction publique française et je voudrais juste dire un mot à mon amie Nicole Duranton lorsqu'elle dit oui, les Allemands, ils font plus que nous, hé oui, mais la haute fonction publique allemande, c'est pas du tout la même chose que la haute fonction publique française. Sommes-nous en manque de hauts fonctionnaires en France de qualité, je ne crois pas combien de préfets sont dorénavant aux Césars, un petit peu être ennuyé, combien de personnes recycle ton parfois à l'IGAS, des anciens ministres très compétent, qui a à l'inspection générale des finances, d'ailleurs, le président de la République lui-même a a dit : je supprime Léna, pourquoi, parce que dans les corps d'inspection, ça serait bien quand même aussi qu'il y ait des gens d'expérience, ben ça tombe bien, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on fait et on ne les utilise pas de lors de la RGPP et ici quelques-uns peuvent s'en souvenir, hé bien c'est simple, on a beaucoup utilisé les corps d'inspection de toutes espèces qui ont certes ne veut jamais eu autant de travail, mais c'était très important, il a même fallu à ce moment-là, une fois que vous avez mobilisé tous ces corps là à voir de temps en temps, un peu d'expérience des cabinets de conseil, alors oui, il faut utiliser la les hauts fonctionnaires, alors certes je comprends que ça plaise pas tellement la ITP qui est telle, la une préfecture, ils avaient les les crédits et puis ils s'aperçoivent que les ministères en font aussi, alors le préfet, c'est la même chose, il s'occupe de représenter l'État sur le territoire, mais en même temps il a pas l'éducation nationale, il a pas la les agences de santé et puis il a pas non plus les ministères des Finances et des ne lui réponde pas non plus, donc, hé bien la DTP c'est exactement la même chose, elle croit centralisé et en fait, il y avait des plein de dépenses de partout, c'est ce qu'a bien révélé la commission d'enquête et donc on voit bien que il y a encore à faire Monsieur le Ministre, je suis sûr que de votre bonne volonté, car je crois que vous, vous avez compris que nous n'étions pas là uniquement pour vous embêter mais pour mieux faire fonctionner l'administration française, je vous ai entendu, j'ai entendu certains de nos collègues, parler des collectivités locales, alors faut quand même pas exagérer hein nous et dans les collectivités locales pour ce con trat qui sont encore élus dans les départements, je ne suis pas sûr que Edgar à nos finances en fasse beaucoup appel au cabinet hein aux honoraires comme cela non puis envisageant lui dire : Monsieur le Ministre, pas vous.

de le de l'administration centrale n'est pas bon sur les cabinets de conseil allait pas donner des conseils aux collectivités locales, commencer par ranger votre chambre avant d'aller voir chez les autres, ça me paraît de bonne politique enfin, un sujet qui est très important pour moi qui est un sujet de souveraineté et de donner, parce que pour moi qui ne savais pourquoi se font-ils payer aussi cher, ils disent : on a des bases de données incroyable et c'est ça aussi qu'on met à disposition, c'est comme ça qu'ils font les les facturations qui oublient de payer les impôts du coup, hé bien ces données, elles sont aux États-Unis, et du coup les lois américaines s'applique sur des données et y compris des données françaises qui peuvent être sensibles et quoi qu'on fasse, on ne peut pas les surveiller alors juste un mot pour terminer, je crois que, avec cette proposition de loi, comme dirait le président de la République, l'abondance est terminé pour les cabinets de conseil. Très bien, merci, la parole est à monsieur Mickael Vallet pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, c'est le président de la commission madame la rapporteure mon camarade Jean-Pierre Sueur vous aurez exposé la position du groupe socialiste, sur les grandes lignes du texte, je me concentrerai pour ma part sur l'article 7 qui impose au cabinet conseil travaillant pour l'État, de bien vouloir, s'il vous plaît, employé la langue française dans les échanges avec l'administration et dans la rédaction de leurs documents, cet article est issu d'une des recommandations de cette commission d'enquête où j'ai siégé avec plaisir et grâce à laquelle nous avons pu mesurer ce qui se passe dans les coulisses de ces marchés publics ou diapositives après diapositives, les cabinets offrent les solutions adéquates que ne saurait trouver par elles-mêmes les administrations. J'aurais pu dire pour me faire mieux comprendre de l'écosystème qui nous occupe et qui nous écoute, peut être que j'ai fait partie du board de la commission qui a mesuré behind comment cela et, d'après slides les consultants juniors et seniors d'un même practices font des propals pour offrir les bon feedback et les qui Learning à leurs prospects public chers collègues si comme moi vous n'entendez rien à ce sabir, rassurez-vous, la commission d'enquête, je vous remercie, Éliane Assassi a annexée au rapport un glossaire du vocabulaire dans les cabinets conseils inondent leurs clients mais inquiétez-vous et inquiétons-nous de la situation qui a rendu ce glossaire malheureusement indispensable. Lors de son audition, le PDG de La Poste, a déclaré que le recours trop systématique au cabinet faisait courir le risque, je cite, d'un nouveau conformisme ce conformisme passe par la langue et conduit à un appauvrissement de la pensée. Ce globish qui n'est même pas de l'anglais est en fait un instrument de formatage, nombreux sont les fonctionnaires et les citoyens, ils l'ont dit à en concevoir une souffrance certaines. La France a un rapport particulier à la puissance publique et à l'administration qui lui est propre, villers-cotterets n'est pas Wall Street et ce rapport entre la France et son administration ne peut être appréhendé par les seuls cabre de pensée outre-Atlantique, ceux-ci correspondent parfaitement la culture anglo-saxonne et c'est une grande culture, mais ce n'est pas la nôtre, et elle ne permet pas de développer souverainement notre propre vision de l'action publique, la légère modification de la loi Toubon proposées dans ce texte ne saurait être résumée à une approche passéiste consistant à regretter le bon vieux temps de l'imparfait du subjonctif, ou de la marine à voile, ce n'est pas non plus la recherche d'une langue pure car une langue figée, est une langue fini, c'est un fantasme morbide que je laisse aux réactionnaires, on doit accepter l'intégration et même avec gourmandise de mots étrangers ou nouveau lorsqu'il recouvre mieux que n'importe quel autre une réalité que notre langue parfois ne décrit pas, en revanche, lorsque le mot existe en français et, surtout, j'arrive au point essentiel lorsqu'il est parfaitement entendu de tous les citoyens, il doit être employé pour que les gens se comprennent entre eux, c'est un impératif démocratique autant qu'un refus de l'entre-soi, une récente étude du Crédoc sur le sujet, rappelle je cite cet attachement manifesté à la langue qui se décline à travers l'expression de la nécessité de service public exemplaire sur le sujet, c'est ce qu'exprime l'article 7 de la présente proposition de loi dans un contexte où les gouvernements de longue date ne respecte ni la loi Toubon ni les dispositions réglementaires prises en application de celle-ci, ni les circulaires primo-ministériel qui s'impose à l'administration les tschüss France French Tech Business France France Connect French Start-Up née Sean bottom up et autres clusters sont autant d'agressions, creusant le fossé entre le peuple et ses représentants, il faut en avoir conscience, quand on est payé par le contribuable, on le sert dans sa langue, ça vaut pour l'administration, comme pour ses dirigeants, comme pour ses prestataires en février dernier, l'Académie française a publié un rapport sous-titré pour que les institutions françaises parlent français, on en est rendu là tout de même en juin dernier le ministre québécois, la langue française en visite à Paris nous inviter avec émotion à ne pas laisser son gouvernement seul dans la bataille, nous devons les entendre, nous avons une occasion rare de renforcer utilement la loi Toubon, Monsieur le Ministre, saisissons-là, d'aucuns inscrivez sur leur slide de conclusion que c'est Nao en never pour réaffirmer les principes linguistique mais avec l'audace dont nous savons faire preuve au Sénat et sur tous les bancs et beaucoup plus clairement, nous pouvons dire que c'est maintenant ou jamais, je vous remercie. Merci, cher collègue, et le dernier orateur, monsieur Stéphane Sautarel pour les républicains. Et également pour quatre minutes. C'est le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, je veux d'abord saluer l'initiative des auteurs de cette PPL Éliane Assassi Arnaud Bazin, dont on a pu mesurer la nécessité lors de la commission d'enquête relative à l'influence des cabinets de conseils sur les politiques publiques, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, c'est donc avec la conviction de la nécessité de cet encadrement que j'ai cosigné cette PPL pour laquelle je vous salue également le travail de la rapporteure Cécile Cukierman. Je ne vais pas développer ici les risques que l'emprise des cabinets conseil peut faire peser sur la démocratie et la légitimité des responsables publics chacun les connaît désormais à un moment de fatigue démocratique forte que connaît notre pays, à un moment où la confiance est pour le moins distendus entre les pouvoirs publics et les concitoyens il convient en effet de compléter notre arsenal législatif pour encadrer ces pratiques en définir le périmètre en piloter l'intervention la robe transparente en encadrer les pratiques et protéger les données de l'administration, je vais me borner ici dans le temps qui m'est imparti à aborder 2 aspects de ce texte, l'interdiction des prestations gratuites qui a déjà abordé, Arnaud Bazin et la protection des données, j'avais beaucoup insisté lors des auditions, comme lors du rendu du rapport de la commission d'enquête sur ce point majeur aussi pro Bono, ses prestations dénuées de tout fondement juridique peuvent répondre à une stratégie du pied dans la porte, visant à développer un réseau d'influence auprès des décideurs politiques et de l'administration, voire à orienter des politiques publiques, je me réjouis que le texte pose le principe de l'interdiction de prestations à titre gratuit : l'équilibre proposé qui vise à autoriser des missions réalisées dans le cas du mécénat d'entreprise au profit de certains organismes ou Oeuvres d'intérêt général, me semble bon il conviendra bien sûr d'un évaluer la mise en oeuvre et la portée pour s'assurer à la fois, qui n'est pas de dérive et que ces organismes d'intérêt général ne soit pas par ailleurs privé de cette ressource, le 2ème aspect que je veux souligner concerne la protection des données de l'administration, s'il est essentiel d'éviter toute confusion entre le consultant et l'administration de l'action publique, comme le prévoit le texte, il est tout aussi essentiel de s'assurer que les données de l'administration utilisés par les cabinets conseils soient protégés, il s'agit bien sûr d'une utilisation pour une finalité autre que l'exécution de la mission confiée à la CNIL, sans obligation d'aviser le prestataire avant une éventuelle vérification sur place, le contrôle de cette suppression de toutes les données ma Paris une mesure équilibré comme la hache TVP mobilisés pour éviter tout conflit d'intérêt, le recours à la CNIL, possiblement autorisée par le juge de la détention des libertés me semble relever d'un bon usage de nos autorités indépendantes. Cette PPL exemplaire en témoignent, les nombreuses réactions du gouvernement suite à la commission de contrôle dont une circulaire insuffisante de janvier 2022, qui a été déjà cité comprend bien d'autres volets qui vont faire avancer nos pratiques démocratiques grâce à l'action du Parlement l'examen détaillé permettra de souligner, chacune de ces avancées dont je me réjouis par avance, notamment en matière de transparence et de proportionnalité, éclairer les décisions oui et nous avons besoin, plus que jamais, de dialogue et d'expertise pour le faire avant, afin de s'accorder sur le diagnostic avant d'engager l'action orienter les décisions par des priorisation de scénario bâti par les cabinets, au travers de chemin près balisé, non, nous ne devons pas être nous non plus des dépossédés comme certains le sont dans cette société, aujourd'hui, je vous remercie pour votre attention et je vous encourage bien sûr à accompagner les débats et a voté cette PPL merci beaucoup. Et nous passons la discussion du texte, la commission, commençons par l'article 1er et Madame Müller Bronn a demandé la parole. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je souhaite remercier mes collègues pour le travail remarquable et inédit, qu'ils ont accompli la commission d'enquête du Sénat a permis de révéler l'omniprésence des cabinets de conseil au coeur de l'État et leur influence sur des décisions stratégiques, notamment dans des domaines régaliens. à ce propos, j'avais déposé des amendements visant à exclure la dimension stratégique des prestations de conseil pour prévenir l'affaiblissement de l'État, l'abandon de sa souveraineté et de ses compétences, j'ai bien conscience des difficultés rédactionnelle et technique qu'ils engendrent, et j'accepte leur retrait. Il faut le souligner, de plus en plus la vie quotidienne des Français est envahie par des recommandations de cabinets de conseil internationaux qui uniformise les mêmes stratégies partout dans le monde, dans les domaines aussi importants que ceux de la santé, de l'éducation, de la justice ou de l'énergie, à titre d'exemple, l'omniprésence du cabinet McKinsey pendant la crise sanitaire illustre l'ensemble des dérives que cette proposition de loi devra encadrer, qu'il s'agisse du confinement des tests PCR des campagnes vaccinales des aides Covid McKinsey a piloté toutes les étapes de la stratégie sanitaire d'autres pays ont décliné les mêmes politiques et on appliqué les mêmes scénarios recommandé par ce cabinet, il serait urgent de stopper la stratégie du copier/coller qui finalement nous entraîne de crise en crise, il serait urgent de stopper la déresponsabilisation des décideurs, il serait enfin urgent de retrouver une stratégie qui relève du courage politique et des intérêts de notre pays. Merci. Nous commençons par l'amendement numéro 19 présenté par Madame Durand, donc il y a la parole. Merci monsieur le président, cet amendement prévoit l'instauration d'un seuil à partir duquel les établissements publics de l'État entreraient dans le Champ d'application de la loi, nous jugeons en effet nécessaire de ne pas faire peser une charge déraisonnable sur des entités de taille réduite, pour lequel les enjeux sont limités, parmi ces entités figurent notamment les chambres départementales d'agriculture, la majorité des Crous, certaines écoles de formation de la fonction publique, certains musées de taille réduite, ainsi que certains établissements publics fonciers concrètement, nous proposons de limiter l'application de la loi aux établissements publics, dont les dépenses donc de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros, ce seuil correspond à celui des avances obligatoire versée aux PME dans le cadre d'un marché public, pour certains, certains établissements publics de l'État avec ce seuil, seuls les plus gros établissements publics de l'État rentreraient dans le Champ d'application de la loi, je pense notamment à la CNAM à Voies navigables de France, à l'Union des groupements d'achats publics ainsi météo France, notre amendement prévoit également la suite. Suppression de l'alinéa IV qui est et répondent qui répondant avec l'alinéa 2 les établissements publics de santé sont en effet une catégorie d'établissements publics de l'État. Merci, la parole à Madame, la rapporteure. Oui merci, bien évidemment, ce sera comme je l'ai laissé entendre dans mon propos liminaire un avis défavorable, non pas parce que, à la question, je l'ai dit du seuil serait devrait être balayée d'un d'un revers de manche tout d'abord, vous l'avez dit, nous pouvons citer un certain nombre d'établissements si ce seuil a été retenu, mais pour beaucoup d'autres, nous n'arrivons pas encore, et ce qu'elles n'ont pas les éléments. Suffisant, les chiffres consolidés pour savoir réellement quels établissements entrerait ou non dans le Champ de la l'application de cette proposition de loi si nous retenons retournions ce seuil des 60 millions et j'entends l'argument que vous pouvez donner, qui est certes un seuil connu encore faudrait-il pouvoir l'expertiser pour connaître la pertinence dans l'application. De cette proposition de loi et donc, comme je l'ai déjà dit en commission, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, ce sera un avis défavorable, parce que la, la commission n'a pas souhaité, en l'état, retenir de seuil. Monsieur le Ministre. davantage logistique de réintégrer l'établissement public de santé dans les établissements publics, puisqu'ils en sont, pour porter sur le 2ème point l'amendement qui vise à fixer un seuil qui dans mon sens, va dans le bon sens puisqu'il va dans le sens de l'effectivité, la proportionnalité de la loi qui est portée, je pense que ça permettra de concentrer l'application de la loi sur les établissements à la fois, qui sont les plus exposés aux risques et à la prévention qu'on doit avoir sur le risque de conflit d'intérêt, mais aussi ceux-là mêmes qui sont les plus à même d'intégrer la contrainte administrative qui va avec la proposition de loi, je crois que ça n'enlèvera pas dans les établissements publics concernés les établissements qui sont visés, je pense à Lucas à l'UGAP, évidemment, vous l'avez mentionné, je pense à Pôle emploi, je pense à des universités, je pense au plus gros établissements publics de santé, je veux dire ici que ça représentera les 500 plus gros établissements public je crois que c'est là l'enjeu et la visée de la proposition de loi et donc je veux affirmer ma position favorable s'installe. Que pu vous demandiez la parole. Pardon, c'est une erreur, donc je mets aux voix l'amendement 19. Pardon monsieur Bazin demande la parole, explications de vote il là.

Un établissement qui brassent des sommes considérables ou un établissement plus modestes, il doit absolument se garantir de tout conflit d'intérêts, je ne vois vraiment pas ce que le la notion de sud faire il vient faire là-dedans, enfin, chiffre d'affaires ou de budget de fonctionnement, si vous préférez donc le la version de la commission, me paraît tout à fait raisonnable, ensuite on verra comment fonctionne tout ça encore une fois, c'est pas du tout une affaire de recettes et de dépenses de fonctionnement, mais bel et bien une affaire de déontologie de prévention des cons, des conflits d'intérêts qui sont, en effet, le cancer de la vie publique, comme l'a rappelé Nathalie Goulet, il faut que ce intransigeant et on ne peut pas, d'emblée, réduire la portée et l'ambition de cette PPL dès le premier amendement, je ne voterai donc pas cet amendement. d'évincer de contraintes déontologiques, un certain nombre d'établissements publics, mais simplement de façon extrêmement réaliste la proposition de loi. Porte un certain nombre de contraintes administratives qui sont tout à fait fondée Jean soutiendrait l'immense majorité dans cette proposition de loi et simplement pour que cette loi soit effective, il faut qu'il y ait une proportionnalité dans les contraintes que peuvent absorber les établissements publics et je pense qu'à juste titre la sénatrice Duranton mentionné un certain nombre d'établissements publics dont on voit qu'il serait en grande difficulté très opérationnel, tout simplement pour appliquer ce que vous proposez donc cet amendement devient à mon sens pas amoindrir la portée, la proposition de loi mais au contraire la renforcer, je voulais clarifier cette police. La présidente, associée à la parole. Oui, merci, merci Monsieur le Président,

la portée et donc l'ambition de notre proposition de loi et je voudrais quand même rappeler que ce seuil de 60 millions d'euros n'a aucune cohérence, en fait, il existe dans le code de la commande publique, mais pour tout à fait autre chose, c'est-à-dire pour le versement des avances donc sur le fond comme la comme cela a été dit par le président Bazin on ne connaît pas la liste des établissements publics qui seraient exclus donc de cette PPL, on peut quand même citer l'institut national du service public, c'est-à-dire l'ex-ENA, l'École nationale de la magistrature l'ENM et certaines agences de l'eau ou certaines agences régionales de santé, donc nous préférons la clarté du texte de la commission et je crois que la PPL doit concerner tous les établissements publics de l'État pour éviter justement les effets de seuil. Je mets le voie d'amendement 19 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement, quels sont ceux qui sont pour.

en mentionnant explicitement qu'elle s'applique à la Caisse des dépôts et consignations, qui comme vous le savez, n'a ni le statut d'établissement public de l'État, ni autoroutier administratives au public indépendante. Avis de la commission madame la rapporteure. cependant elle faisait bien partie du travaux de du périmètre des travaux de la commission d'enquête et donc pour ces raisons-là, ce sera un avis favorable. J'émettrai pour ma part, un avis de sagesse, monsieur le président, effectivement, la Caisse des dépôts, c'est un établissement par, effectivement, il fait déjà l'objet d'un contrôle parlementaire, puisque sa commission de surveillance est présidé par un parlementaire, en l'occurrence, qu'on pourrait envisager, effectivement, le fait que ce contrôle soit déjà existants qu'puisse être considéré un peu à part, mais je préfère émettre un avis de sagesse si la Haute assemblée souhaite l'intégrer dans le périmètre de la proposition de loi.

et non pas la Caisse des dépôts seulement typiquement lors de la commission d'enquête, nous avons entendu Philippe Val, le PDG de La Poste qui est dorénavant, filiale de la Caisse des dépôts, avec le contrôle exclusif et c'est notamment tout cela parce que la Caisse des dépôts, c'est bien mais c'est dorénavant le groupe que des dépôts ou la Caisse des dépôts et ses filiales, comme dit le le texte donc moyennant cela, ça pourrait être corrigé dans une navette car vous ne manquerez pas monsieur le ministre de l'inscrire à l'Assemblée nationale. Je mets aux voix ah pardon. Nous, on a eu les avis. Donc je mets aux voix l'amendement 27 avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre, il est adopté, nous avons ensuite 4 amendements en discussion commune, commençons par le 1er rectifier

je veux le redire à une force, il lui reste simplement un écueil que je vous propose de corriger ça va tendre pour la suite, dans la navette, une partie de l'administration publique a été oublié, comme l'état de collectivité prenne des décisions politiques qui aime pas que la vie, nos concitoyens, et comme l'étage susceptibles de faire appel à des consultants, engageant ainsi les finances publiques, aussi, il n'apparaît pas tout à fait absurde de vouloir mieux encadrer ces recours même si nous savons qu'il existe déjà des mécanismes permettant que ce soit par le biais des cours régionales des comptes ou du contrôle par l'opposition,

cet amendement propose donc d'inclure dans le périmètre de cette loi, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à la terrifiante des communes de moins de 10000 habitants, ainsi que les intercommunalité à l'exception des communautés de communes, était trop bas aussi ils ont également déposé un amendement de repli qui est le numéro 45 de repli qui retient comme limite 100000 habitants et ainsi que l'intercommunalité, à l'exception des communautés de communes. Merci président ensuite le second amendement en discussion commune monsieur le projet de loi. Doit. Correspondent exactement au périmètre de la commission d'enquête. Ils disent : on ne peut pas aller au-delà. Mais je ne comprends pas pourquoi. Nous sommes des législateurs, nous pouvons déposer des amendements et si nous trouvons qu'on peut élargir le Champ qu'il faut le faire, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. C'est pourquoi nous proposons par cet amendement de d'étendre les bienfaits de cette loi aux collectivités locales, avec un seuil qui est différent de celui présenté par notre collègue et ami Monsieur Ruquier dans son premier amendement mais conforme à celui du second amendement, c'est-à-dire qu'il nous paraît sage d'exclure les communes de moins de 100000 habitants mais d'appliquer les règles qui sont fixées dans le texte aux communes de plus de 100000 habitants aux autres collectivités locales et aux intercommunalités de plus de 100000 habitants. Le 45 a été présenté par Monsieur Ruquier et donc il nous reste le quarante-quatre présenté par le gouvernent. Oui, monsieur le président, mon argumentation sera assez similaire à celle qui vient d'être porté par le questeur sueur et président Ruquier, au fond, elle repose sur l'appréciation même qu'on a de la proposition de loi, soit on considère que cette proposition de loi est punitive pour la puissance publique qui s'applique, je crois que ça n'est pas votre cas et ça n'est pas mon cas, ce soir, soit on considère que les dispositions qui sont portées dans la proposition de loi sont des dispositions qui viennent renforcer les acteurs publics qui sont concernés, et à ce moment-là je vois effectivement pas de bonnes raisons de ne pas inclure dans le Champ de bénéfice des dispositions qui sont dans cette proposition de loi, les collectivités territoriales, je crois qu'il y a pas de débat et si ce soir, sur le fait que les collectivités terrain. Territoriales ont recours à des organismes de conseil, ça peut être une région qui a recours parfois pour quelques centaines de milliers d'euros quand il s'agit de bâtir la politique stratégique d'attractivité économique, ça peut être parfois un département qui a recours à des missions pour quelques dizaines de milliers d'euros quand il s'agit de bâtir le schéma directeur en matière de politique sociale, ça peut être parfois une collectivité une métropole quand il s'agit de réorganiser des services, je prends la des exemples sont des exemples concrets effectif de la vraie vie de ces différentes collectivités et donc je considère comme certains ici et sur différents bancs de l'Assemblée, que l'intégration des collectivités et pas punitive à à leur égard, mais au contraire permet d'étendre le Champ de la loi et de leur en faire bénéficier sur la question du seul, je crois, effectivement vous m'entendrez souvent parlé de personnalité : ce soir, mais que il y a une bonne forme de proportionnalité, a considéré que les collectivités au-dessus de 100000 habitants, c'est-à-dire les régions, les départements, les 42 communes communes les plus importantes soient concernés à la fois parce que elles ont de la même façon que sur l'amendement précédent la capacité à intégrer les contraintes administratives pour pouvoir répondre et se mettre en conformité avec les dispositions de la PPL et parce que je crois qu'elle a un Champ prioritaire pour regarder si il y a effectivement vocation à les protéger de conflit d'intérêt, c'est la raison pour laquelle, pour ma part et au nom du gouvernement j'ai déposé un amendement à 100000 qui est d'une écriture, un tout petit peu différente par rapport aux amendements qui ont été déposées, considérant que les EPCI de plus de 100000 habitants doivent être pris en compte et pas toutes tailles de PCI c'est la seule différence entre les amendements qu'on a pu déposer. Alors l'avis de la commission sur les quatre amendements madame la rapporteure. Bien, comme je l'ai également déjà dit la discussion sur les collectivités territoriales et légitime, donc la question n'est certainement pas de balayer très trop rapidement ce débat là, cependant je veux également dire, puisque chacun pose des préalables, mon collègue Jean-Pierre Sueur que personne ne dit que la loi ne peut pas aller plus loin, en revanche, je vous ai proposé, en concertation avec les auteurs en commission des lois, un équilibre politique qui respecte effectivement l'accord tels que sorti de la commission d'enquête et qui rassemble l'ensemble des auteurs de cette proposition de loi qui est hein. Point d'équilibre et qui vise, en tout cas, lors de cette première lecture ici au Sénat, à ne pas trop déroger et ne pas aller sur des champs qui n'ont été ni à investiguer par la commission d'enquête ni investiguer, j'oserais dire humblement par la rapporteur de la commission que que je suis ensuite je, je, je souhaite dire également le faire remarquer, peut-être avec un peu d'ironie, vu l'heure tardive, qu'il y a, effectivement, c'est un vrai sujet, il y a 4 amendements avec des rédactions différentes, avec des seuils différents avec des collectivités ou en tout cas leurs groupements qui ne sont pas toujours les mêmes, j'oserais dire, preuve en est : si, si, il y en avait besoin que cela demande un peu de temps un peu d'expertise pour être au plus juste et puis enfin, et parce que nous sommes ici au Sénat, je veux notamment attirer l'attention tout d'abord de mes collègues qui ont déposé de tels amendements mais également, là encore, avec humilité, monsieur le Ministre de de vous-même, je crois que, à l'heure où demande beaucoup de concertation à l'heure où nous voulons construire en partant de la réalité des territoriales construire en partant de la réalité vécue par les élus locaux, qu'il serait malvenu, mais surtout peu efficace, peu opérationnel de faire entrer les collectivités territoriales, par la voix de tels amendements sans même s'interroger, y compris sur les conséquences que cela aurait sur un certain nombre d'articles ou sur un certain nombre en tout cas de mesures prévues par les autres articles pour les administrations de l'État et qui donc de fait ne rendrait pas effective l'application de cette proposition de loi aux collectivités territoriales, et donc nous proposons plutôt de pouvoir effectivement menées mission commission d'enquête, bref, quel qu'en soit la situation, en tout cas de travailler en profondeur avec les élus locaux, les représentations des associations de collectivités territoriales céderait question de l'utilisation, s'il y en a excessive des cabinets de concernant les collectivités territoriales et des règles de déontologie qu'elles doivent s'appliquer qu'elles doivent mettre en oeuvre et qui seront inévitablement différente à certains degrés que celle que l'on peut attendre et mettre en place pour les administrations de l'État.

vous avez évoqué 2 arguments au fond que je voudrais répondre : le fait que, il y aurait un travail à mener pour parfaire les dispositions qui serait encore devant nous, vous avez-vous qu'un 2ème, argument qui est de dire au fond qu'on mesure mal l'impact réglementaire financier sur les collectivités, des dispositions qui sont prises dans le texte, je veux évoquer de contre-arguments sur l'étude d'impact et sur l'impact qui aurait lieu sur les collectivités, vous n'avez pas eu ces réserves là sur les établissements publics de santé. Il y a 220 hôpitaux locaux dans le texte de mémoire 3300 établissements publics de santé qui sont concernés, je ne crois pas que la commission d'enquête sénatoriale se soit penché sur les conséquences, vous avez auditionné, Martin Hirsch, je crois que c'était effectivement la seule audition qui a été menée pour pouvoir évoquer les conséquences sur les établissements publics de santé et aujourd'hui vous évoquez cet argument pour dire au fond, on n'a pas pu le faire pour les collectivités et puis vous avez dit vous-même madame la rapporteure, le texte n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ, c'est-à-dire qu'il y aura une navette parlementaire, on avait parlé à plusieurs reprises ce soir j'ai indiqué que je souhaitais que le texte puisse cheminer et donc il est tout à fait possible dans le temps de la navette parlementaire de pouvoir travailler et je veux le dire devant vous, je suis extrêmement ouvert sur la forme, vous avez évoqué le fait de nommer des parlementaires en mission pour pouvoir avancer sur ces questions là, moi je suis prêt à le faire et à donner les moyens à l'assemblée de le faire dans le cadre de la navette parlementaire pour pouvoir effectivement par faire le texte envoie exactement les conséquences concrètes, donc vous voyez que j'ai une position très sincère face à vous pour défendre cette position d'intégrer les collectivités à ce stade du texte qui, je vous cite, est un point de départ. Qui veut dire que vous êtes favorable trois amendements. Je suis favorable à l'amendement présenté par le gouvernement pour les raisons évoquées, je propose le retrait des 2 amendements similaires, en tout cas sur les seuils qui ont été déposées pour la raison que j'évoquais tout à l'heure de cohérence par rapport aux EPCI si le seuil est au-dessus de cent je propose qu'il soit aussi 200000 pour toute ta de collectivités et c'est inclus dans l'amendement quarante-quatre de mémoire du gouvernement et donc je vous propose de retenir cette rédaction là donc, proposition de retrait pour les 2 précédents et avis favorable évidemment sur l'amendement gouvernemental. D'abord, Monsieur Richard souhaite expliquer son vote. C'est le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai été de ceux qui, en réunion de la commission des lois se sont émus de l'absence des collectivités locales dans le périmètre d'intervention de ce texte et je dois dire que je me suis interrogé sur la possibilité de présenter un amendement j'ai un peu travaillé et je dois dire que j'ai été excusez-moi le terme, j'étais sec devant ma feuille blanche,

j'aurais pu penser à l'Alsace, parce que c'est plus proche de moi, enfin cette région que j'espère retrouver bientôt d'ailleurs à la place du Grand-Est, mais c'est un autre débat, mais l'autre, l'autre entrée c'était naturellement le seuil et le seuil j'ai j'ai vu Jean-Claude Requier m'excusera mais on passe de 10000 à à 100000 on sait pas pourquoi Jean-Claude c'est bon, ça pouvait être cinquante mille ça vaut une 20000 c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que les conséquences sont quand même relativement lourde pour les collectivités concernées et donc franchement, j'ai été convaincu par les explications qui m'ont été donnés par Madame la rapporteure en commission répéter ce soir, il faut vraiment mener un travail approfondi sur ce dossier, il n'a pas été menée, quelles que soient les formes qui pourraient être celles de cette concertation nécessaire dans le cadre de ce travail approfondi, il me paraît indispensable que celle-ci ait lieu, deuxièmement, moi je suis vraiment très sensible à l'observation tout à l'heure de le président de la Commission, monsieur Bazin je crois que la question de la déontologie l'emporte sur la question du seuil, nous avons tous en tête en tête l'un ou l'autre cas d'espèce dans certaines collectivités qu'il vaut mieux ne pas citer par ce soir, qui amène à se poser des questions en termes de tellement de déontologie indépendamment du seuil et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut faire un travail approfondi sur ce dossier, moi, je voterai contre cette extension aujourd'hui mais je répète, il faudra faire ce travail et et se prendre le temps pour le faire monsieur le président, Monsieur le Ministre, en effet, la question est légitime et c'est une des premières questions que nous nous sommes posés avec Éliane Assassi après la fin des travaux de la commission d'enquête pour savoir ce que nous allions retenir dans la proposition de loi dont nous débattons ce soir nous est assez vite apparu qu'il ne fallait pas inclure les collectivités territoriales pour les raisons qu'a rappelé la rapporteure, mais je voudrais insister sur 2 points qui sont à mon sens tout à fait déterminant le 1er point, c'est que l'influence des cabinets de conseils sur l'état concerne à l'évidence des sujets beaucoup plus vaste, y compris dans le domaine de la défense nationale ou dans le domaine sanitaire elles intéressent toute la nation, tandis que les décisions prises dans un département ou d'une dans une région si elles ne sont pas négligeables sont quand même beaucoup plus limités dans leurs conséquences. Et puis, surtout, surtout, pourquoi est-ce que nous sommes là parce que nous avons constaté qu'il est nécessaire de renforcer la transparence, on a dit transparence, contrôle du recours déontologie mais le 1er point, c'est la transparence et il nous a fallu tous les outils d'une commission d'enquête avec tous ses pouvoirs, qui ne sont pas minces audition sous serment communication obligatoire des documents vérifications sur place et sur pièces pour savoir ce que le de l'État dépenser en matière de cabinets de conseil de consultants, il nous a fallu tout ça donc pour avoir notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement, il nous a fallu toute tous ses moyens, nous avons prévu de les entrées de les faire entrer dans la loi, mais que se passe-t-il dans les collectivités territoriales, il y a des assemblées délibérantes il y a des oppositions, il y a des communications obligatoire de documents quand j'étais président du département du Val Oise j'ai fourni à mon opposition tout un ensemble de documents et ils ont le le compte administratif, les comptes de gestion par ailleurs et puis il y a aussi l'encadrement par les services de l'État par la trésorerie qui vérifie que les décisions sont conformes à ce qui a été votée, donc il y a tout un appareil tout un contre-pouvoir qui est déjà en place dans les collectivités locales, ça n'empêchera pas de se pencher sur le sujet, mais je veux dire que les choses sont absolument pas symétriques absolument pas comparables, c'est pourquoi nous avons choisi de ne pas retenir les collectivités territoriales. Ensuite, madame Assassi. sur Monsieur le Ministre, les décisions de l'état de ces établissements publics et de CV et des hôpitaux. Nous avons aussi intégrer les hôpitaux dans les travaux de notre commission d'enquête sur les collectivités aujourd'hui parce que j'entends bien évidemment les amendements qui sont déposés par nos collègues et je pense qu'il ne faut pas être sur la défensive sur sur le sujet, il faut savoir l'aborder frontalement et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons été plusieurs à émettre l'idée que le Monsieur le Ministre, puissent rencontrer les associations d'élus pour avoir un échange approfondi avec elle sur ce sujet que ce puis sans doute peut-être faire l'objet d'un d'un rapport, on a parlé, je crois que c'est Madame rouler tout à l'heure qui proposé, pourquoi pas une mission flash mais des parlementaires pourraient aussi demander une commission, une mission d'information, une commission d'enquête sur le sujet parce que c'est un vrai sujet, on ne se le cache pas, il y a des collectivités parmi les plus importantes qui effectivement ont recours à des cabinets privés mais aujourd'hui nous n'avons aucune donnée consolidées sur le niveau des dépenses de conseil des collectivités territoriales, puis Monsieur le Ministre, excusez-moi, mais il y a quand même un paradoxe à vous voir très disposé pour étendre la PPL aux collectivités, alors que vous avez déposé plusieurs amendements pour réduire l'ambition de notre texte sur ses propres services. Et enfin Madame Gatel. à mon tour me réjouir du travail qui a été conduit par les présidents à ceci et Bazin je trouve que ça illustre parfaitement la capacité du Sénat à dépasser les clivages à prendre le temps de travailler sur le fond, sur des vraies questions et des sujets importants, monsieur le ministre, moi je partage la nécessité pour l'État, comme pour les collectivités de recourir à des expertises extérieures et en tout cas, il n'est pas dans l'intention du groupe centriste pratiquer une sorte de chasse aux sorcières, maintenant, nous sommes tous d'accord sur la nécessité de plus de transparence, d'exigence et de contrôle, monsieur le Ministre, vous avez raison, se pose la question des collectivités, il ne faudrait pas que quelqu'un en nous écoutant ce soir et l'impression que nous, nous dérouillons et que nous voulons échapper à la transparence, c'est pas le genre de la maison et autre chambre voilà mais Monsieur le Ministre, vous avez salué la qualité, la rigueur du travail qui a été fait, la qualité et la rigueur conduisent à avoir eu une expertise, une évaluation, faire des propositions maintenant la la mission, elle a écarté de son Champ de travail, les collectivités, maintenant, vous voyez bien que nous disons tous qu'il y a un champ investiguer mais pardonnez-nous, nous n'allons pas décidée à la hussarde, à 24 heures enfin même un un peu plus de ce qu'il va arriver aux collectivités, alors même que nous ne les avons pas entendu et que nous ne cessons vous comme nous, y compris le président de la République et les collectivités de déplorer le fait qu'il peut arriver à quelqu'un, prendre une décision sur un coin de table ou au coin d'un d'un fauteuil d'imposer dit zut, ça marche pas, donc Monsieur le Ministre, d'ailleurs, si je puis me permettre sans malice : je me demande pourquoi sur votre amendement, il manque les métropoles de Marseille et de Paris, qui ont un statut particulier, mais peut être et je m'allume la la, à votre proposition et qu'on voit bien qu'on a un éventail de propositions qui nécessite, Monsieur le Ministre, avec sérieux et avec exigence d'aller investiguer mais ce soir, je pense que vous seriez le 1er à regretter ce que nous pourrions faire parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc que la mission soit poursuivie ici ou que l'Assemblée nationale prenne le sujet, moi je suis OK mais sincèrement, on ne peut pas décider d'un truc comme ça, le sans en avoir parlé aux associations d'élus, merci monsieur le président.

il faut dire que j'ai pu constater des des dérives en matière de recours à des cabinets conseil et je fais un pas par rapport aux enjeux déontologiques je pars plutôt sur le contenu de de de ce recours parce qu'il est parfois faire recours parce que la loi suscite ce recours à des cabinets de conseil à travers des exigences tels que l'érable de rations d'un certain nombre de documents stratégiques de développement ou autre, à travers des documents du d'urbanisme et que cela peut avoir des conséquences particulières : tout d'abord la standardisation des des approches sur la manière d'aborder les sujets, on a des formes que copier/coller, alors sinon matériel au moins à un moment où il nous faut repenser l'ensemble des concepts l'ensemble des compromis sur les différents enjeux de société également et évoqué souvent par rapport à des documents ou en tout cas des, des, des, des schémas qui ne sont, comment exiger une absence parfois une insuffisance de maîtrise des travaux par les fonctionnaires de la collectivité territoriale, parfois par les élus qui conduit à une forme entre guillemets de délégation de pouvoir, il s'agit, à travers effectivement ce regard sur l'intervention des cabinets conseil de s'assurer que, on n'a pas cette facilité du recours aux cabinets que et conseils et que ce soit effectivement réservée, là où il est nécessaire d'avoir des expertises en particulier techniques nécessaires pour pouvoir mener et définir les politiques locales Françoise Gatel tout à fait légitimement et ce que j'avais annoncé à la tribune d'une double sincérité très centriste, nous allons nous abstenir sur l'ensemble de ces, de ces amendements parce qu'effectivement il y a un sujet, donc il est pas question de de voter contre et en même temps, le périmètre de la mission et la nécessité d'avoir des auditions et un travail plus précis, fait qu'on ne peut pas voter pour, donc, nous nous abstiendrons. Bien monsieur capuche. Les discussions que nous avons sont très intéressantes, elle démontre le fait que ce texte est extrêmement complexe, d'un côté on dit la notion de déontologie et tu ne tu n'est pas une notion de chiffre d'affaires ou de budget de fonctionnement, et donc on ne peut pas ne l'appliquer aux établissements publics administratifs de plus de 60 millions d'euros de budget seulement et de l'autre, on dit : ah, on ne peut pas appliquer le sept cet article aux collectivités territoriales, qui ont 100000 habitants, c'est-à-dire un budget de fonctionnement de près de 500000 euros au moins,

à faire le périmètre et qu'il y qu'on dit en fait un peu tout et son contraire sur le même article, c'est la raison pour laquelle il me semble que ce texte n'est pas prêt, c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai madame le rapporteur. Non, simplement sur quelques éléments qui qui ont été apportées, je, je, je pense que jusque-là chacun à éviter de caricaturer les propos des autres il est important que nous puissions d'abord qu'on continue à avancer ainsi donc voilà je, je pense qu'aucun collègue ici n'a dit à aucun moment donné que la question des collectivités territoriales dans n'était pas eu la seule chose sur laquelle je crois plusieurs alertes tout d'abord, notre collègue Arnaud Bazin le rappeler. Précédemment, il existe aujourd'hui des mécanismes, alors je ne sais pas si on doit dire de contrôle de régulation de transparence ou d'information dans les collectivités territoriales qui sont différents de ceux qui sont mis aujourd'hui dans la plupart des administrations de l'État, deuxièmement, cela a été dit par Madame Assassi par Madame Gatel, par un certain nombre d'autres la volonté. Que cette question des collectivités territoriales, notre collègue Richard également ne soit pas simplement entre guillemets, la roue tourne ou correspondant à telle référence à l'article du du code général des collectivités territoriales mais qu'il y ait plus largement. Une une expertise et surtout une réflexion avec celles et ceux qui au quotidien les administre, c'est-à-dire les élus, les élus locaux en situation d'exécutif aujourd'hui et puis mais je le redis, c'est-à-dire parce que je, je viens d'entendre ce qui ce qui ce qui a été dit par notre collègue kaput mais non, aujourd'hui, cette proposition de loi. Si on rentre les collectivités territoriales, effectivement, je serai envie de dire, je pourrais vous avez raison, tout un certain nombre d'articles vont devenir complètement incompréhensible mais par exemple, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de de ce que l'on exige à l'article 8 pour les collectivités territoriales,

Monsieur le Ministre. pour les établissements publics, dont vous avez choisi de ne pas mettre de ce dans l'article 1er en concernant un certain nombre de mesures vous c'était celle de l'article 8 c'est exactement la même question qui va se poser pour certains établissements publics de petite taille, je veux simplement notifié 3 points sur les sujets qui ont été abordés, d'abord sur la question des seuils, je peux comprendre le syndrome de la page blanche, au moment de rédiger, je veux simplement dire que la seuil et la rédaction même que nous avons choisi, c'est l'exact rédaction qui a été adopté par cette assemblée sur la loi de transparence de la vie publique de 2013 exactement la même, donc d'une certaine façon, je voudrais enlever vos préventions sur ce sujet-là 3ème point il me semble, monsieur le président, Bazin qui a un argument qui est quelque peu circulaire, vous dites au fond, il ne faut pas prendre les mesures pour les collectivités, parce que nous n'avons pas une bonne connaissance du recours aujourd'hui par les collectivités au cabinet de conseil mais justement la proposition de loi dans les discussions que nous allons avoir juste après sur les articles 3 4 et 8 permettent de faire plus de transparence en listant les recours aux prestations par les cabinets de conseil et puis dernier point vous dites au fond ce ne sont pas exactement les mêmes enjeux déontologiques pour l'État dans le Champ est plus large que pour un certain nombre de collectivités, c'est l'argument que vous avez mentionné tout à l'heure, cet argument-là, pardon, mais je ne peux pas partager les enjeux des collectivités sont des enjeux de la vie quotidienne des Français sur les questions extrêmement central de logement, d'action sociale de transport, je crois que ce sont des enjeux sur lesquels les enjeux de déontologie sont tout aussi existants, que ce qui concerne l'état et donc c'est la raison pour laquelle je persiste à émettre un amendement un avis favorable sur ces amendements. Je mets aux voix. Mes chers collègues, nous sommes toujours d'accord pour finir cette nuit. Nous sommes à trois quarts d'heure pour ne pas encore avoir examiné 6 amendements. monsieur le président, je voulais vous dire simplement que le seuil de 10000 c'était un 1er le trouver trop bas, on a mis à 100 mille mais je dis pour accélérer les choses que je retire l'amendement numéro un et je retire le numéro 45 au profit du

Qui est contre,

On finit sur l'article 1er n'ont pas encore d'ailleurs avec l'amendement vingt de Madame Duranton. les prestations de conseil en gestion de ressource humaine, nous considérons que ces prestations, à l'instar de l'aide au recrutement ne relève pas du Conseil stratégique mais vient essentiellement à répondre aux besoins pratiques des administrations. Oui, ce sera atteint un avis défavorable puisque, au contraire, il me semble que le projet de restructuration et de transformation, peuvent en effet comprendre un volet relatif aux ressources humaines et de fait. Supprimer les mots et en gestion de ressource humaine serait affaiblir la portée de la loi.

Juste un mot, monsieur le président, Monsieur le Ministre, cet amendement consiste à déplumer considérablement la loi parce qu'il y a beaucoup de recours justement à des cabinets de conseil pour des recrutements, des évaluations pour tout ce qu'on appelle aux ressources humaines et caetera, donc il est essentiel que cela reste dans la loi.

en accompagnement aux ressources humaines et de recrutement d'un analyste opérationnel à Santé publique France qui entrera en fonction le 23 septembre 2020, identification de profil, recueil de CV, prise de contact, proposition de profil, réalisation des entretiens avec esprit, avec Santé publique France matrice de synthèse des candidats short-listés, donc on est vraiment sur des sujets très très délicat et pointus qui engagent des politiques régalienne de l'État, c'est pas du tout neutre. Donc. Je mets aux voix l'amendement de Madame Duranton le vin avec un avis défavorable de la commission, un avis favorable du gouvernement qui est pour.

au sens de la loi, l'article 1er prévoit. Fusion dans la catégorie des consultants, des personnes physiques qui s'engagent à titre individuel avec l'administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil si les termes qui s'engage, renvoie assurément aux personnes physiques ayant passé un contrat avec l'administration bénéficiaires les termes à titre individuel sont quant à eux beaucoup plus ambigu et source de difficultés d'un prix d'interprétation, une lecture extensive de ces termes pourrait par exemple conduire à inclure dans la définition des consultants les agents contractuels de droit public ou les vacataires recrutés pour assurer des tâches ponctuelles relevant des prestations de conseil de tels agents sont en effet des personnes physiques qui s'engagent à titre individuel, avec leur administration d'emploi or il convient de ne pas inclure les ressources humaines internes à l'administration dans le Champ d'application de clarté et d'intelligibilité de la loi, nous proposons de substituer au terme à titre individuel les termes en qualité d'indépendant, les agents de l'administration, recrutés par contrat seraient ainsi clairement exclus du Champ d'application de la loi, alors que les personnes physiques exerçant des activités de consultance au profit d'une administration sans être employée ni par celle-ci, ni par un cabinet de conseil serait quant à elle, soumise au respect de la loi. Avis de la commission s'il vous plaît madame la rapporteure. Oui, ce sera un avis défavorable puisque, là, dans cet article le à titre individuel. Son temps ici par contraste par rapport à ceux qui interviennent au travers d'une personne morale, et donc nous souhaitons on rester à la rédaction, telle que proposée par la commission. Monsieur le Ministre. par l'attaque de loi et j'insiste une seconde sur l'ambiguïté du terme, à titre individuel, ce serait quand même extrêmement dommageable que des agents contractuels rentre dans la définition de la proposition de loi donc j'insiste sur l'avis favorable que pour ma part, je pense, sur cet amendement. Je n'ai pas de demandes de parole donc je mais aux voix l'amendement 21. De madame Duranton, qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement qui est pour.

non, le huit est maintenue, donc vous avez la parole madame. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, alors cet amendement a pour objet de s'assurer que l'expertise sous-traité par l'État aux cabinets de conseil reposent sur de réelles compétences, le rapport de la commission du Sénat, ainsi que l'enquête publiée par 2 journalistes, intitulé Les infiltrés ont révélé le manque de rigueur et le caractère parfois désinvolte et inutile des travaux livrable rendu par les consultants, exemple de la recommandation par McKinsey pour la campagne sur la quatrième dose de vaccination, l'unique scénario porte sur 100 pour 100 d'adhésion, le scénario de réduction des coûts sociaux sur la baisse de 5 euros de l'APL, on voit ce qu'il en reste aujourd'hui ou l'invention des masques grand public qui a été, de la part d'une agence publicitaire une décision publicitaire et non pas une décision d'autorité sanitaire. Merci, oui, de la commission. Oui, tout d'abord, je remercie notre collègue Müller Bronn pour avoir retiré effectivement ces amendements parce que. C'est nous, si nous en avions eux-même la les l'état d'esprit de départ en en tout état de cause, vu les rédactions proposées, ils allaient presque à l'encontre de ceux qui était recherché en revanche j'émettrai là un avis défavorable de la de la Commission puisque cela nous semblait dans un degré de précision qui ne semble pas utile et et pas effectif pour la, pour ce qui est recherché à l'article 1er de cette proposition de loi. loi. Le ministre. Même avis que le rapporteur Monsieur le président, pour la raison très simple, que l'ensemble des prestations de conseil ne repose pas forcément et systématiquement sur des données chiffrées et donc et un problème, à mon avis d'application de cet amendement. Bien.

l'affluence, la lutte contre l'influence des cabinets de conseil sur la décision publique il nous semblait important que ces cabinets de conseil privés indique aux administrations les différentes pistes qui sont envisagées lors de la construction de projets pourquoi c'est en fait pour ne pas laisser une marge de manoeuvre disproportionnée au consultant dans le choix du scénario proposé bien entendu, le choix du scénario reste toujours la responsabilité des consultants, mais le fait de devoir pour un prestataire ou un consultant par principe proposé ou faire état de l'ensemble des scénarios envisagés permet aussi, dans ce cas de motiver la décision d'abandon de la ou de l'autre des scénarios, ce qui nous semble être une garantie supplémentaire. Oui, ce sera un avis défavorable, parce que, à travers cet amendement, même si nous pouvons mesurer le sens il rendrait complètement in opérationnel en pratique l'application de de de cet article 1er en effet, la liste des scénarios n'auront, pourrait devenir illimité. Et donc ainsi prêté quoi voilà prêter des intentions qui ne ne pourrait jamais cessé ni stopper et, de fait, même si la volonté est effectivement d'aller vers plus de transparence, plus de justification dans ce qui est retenu par rapport à ce qui n'est pas retenue telle que rédigée tels que propose proposer cet amendement viserait certainement plus à bloquer qu'à assurer plus de transparence en la matière.

Entre. Tension et il n'est pas adopté Madame Mélanie Vogel nous présente l'amendement 28. Merci monsieur le président, donc, cet amendement vise à créer une incompatibilité légale formelle entre les cabinets de conseil qui contractualisé avec l'État et les cabinets d'affaires publiques qui comptera actualise auprès de clients privés pour exercer en leur nom des activités de représentation d'intérêts auprès des décideurs publics, la mission d'enquête parlementaire, et notamment son audition du président de la Haute autorité, a bien démontré que les cabinets de conseil intervenant auprès de l'État n'étaient pas des représentants d'intérêts au sens propre et n'était donc pas inscrit en tant que telle, au répertoire de la Haute autorité, sauf rares exceptions, mais le risque évidemment sans garantie légale réaffirmé ce serait qu'un cabinet de conseil se prévalent de sa mission auprès de l'État pour vendre auprès de ses clients privés une influence supposée ou réelle, qui constituerait un Avantage indu et pourrait même s'apparenter, dans certains cas un délit pénal de trafic d'influence, il apparaît donc nécessaire et utile d'établir légalement que les cabinets de conseil qui contractualiser que l'État ont l'interdiction d'effectuer toute action de représentation d'intérêts auprès des pouvoirs publics, au nom de tiers et je veux bien sûr préciser que cette interdiction n'exclut pas du tout la possibilité que ces cabinets effectuent des actions de représentation d'intérêts en leur leur propres en leur nom propre ou via leurs associations professionnelles, mais simplement au nom de tiers, je vous remercie. Avis de la commission. pour justement faire de la représentation au profit d'un autre client ce d'un autre client pardon serait de fait en conflit d'intérêt et donc punissable par la Haute autorité la la. Transparence de la vie publique et donc, il ne semble pas opportun d'apporter la précision d'une incompatibilité général entre ces professions.

Et contre. Et il est adopté, après l'article 1er, passons à l'amendement 26 présenté par monsieur que dès lors que les mesures proposées par ce texte sont bénéfiques et nous croyons vraiment qu'elles sont bénéfiques pour l'ensemble des services de l'État. Il est logique que nous puissions aussi les ça les les s'appliquer aux assemblées parlementaires, je trouve que, dès lors qu'il y a une bonne. Série de mesures qui s'appliquerait à l'ensemble des ministères, je ne vois pas pourquoi ces mesures ne s'appliquerait pas non plus aux assemblées parlementaires, je précise qu'il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause l'indépendance des assemblées parlementaires, de même que la loi qui a créé les représentants d'intérêts s'applique au Sénat. Dans les conditions fixées par le bureau du Sénat en toute indépendance, nous proposons dans notre amendement que les dispositions de la présente proposition de loi s'applique au Sénat comme à l'Assemblée, selon les modalités qui seront mises en oeuvre par le bureau de chaque assemblée pour préserver absolument cette indépendance. au bureau des assemblées par parlementaires de mettre en place leurs règles sont base légale que là encore au travers un amendement visait ainsi à imposer par la loi, cette, cette extension j'oserais dire d'application aux Chambres parlementaires nous semble un peu rapide rapide et en tout cas là aussi prématuré, donc l'avis est défavorable. S'il n'y a pas d'observation, je mets aux voix l'amendement 26 du président sueur qui est pour. Qui est contre il est pas adopté, je peux donc mettre aux voix l'article de. Qui est pour. Contre. Claude est adopté, nous passons à l'article 3 sur laquelle ont demandé la parole, la présidente Assassi ensuite monsieur la. Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement est très important car en fait qui l'acte le recul du gouvernement sur la transparence des prestations de conseil, il faut d'ailleurs le replacer dans son contexte, évoqué lors de la discussion générale, nous sommes dans une situation où, par exemple par le journal Le Monde est obligé d'aller devant le tribunal administratif pour obtenir des informations, en pratique, les ministères ne répondent pas aux demandes des journalistes, ils refusent de donner les documents et perdent devant la Cada, mais il joue la montre, ils savent que la procédure judiciaire va prendre des mois voire des années, et qu'il reste tranquille, entre guillemets, pendant ce temps, c'est notamment le cas du rapport McKinsey sur l'avenir du métier d'enseignement, d'enseignants, pardon, que le gouvernement refuse toujours de publier d'une manière générale, nous assistons à un retour de l'opacité, depuis la fin des travaux de la commission d'enquête sous des airs technique cet amendement supprime au moins quatre garanties de transparence prévue par d'autres textes, premièrement, la publication des bons de commande qui sont pourtant communicable selon la Cada pour transmettre ces documents, il suffira donc de biffer le nom du fonctionnaire en charge qui ne me semble pas ce qui me semble très abordable à l'heure du numérique, deuxièmement la cartographie RH des ministères que nous demandons, afin que l'État puisse mieux mobiliser ses compétences internes et moins recourir aux consultants extérieur,

le gouvernement propose un délai de 2 ans et pour l'ensemble des des établissements publics public le gouvernement souhaitant décentraliser la formation de chaque établissement et ainsi la rendre par les établissements publics sont certes autonome sur le plan administratif mais sont surtout rattaché à une ministère de tutelle et donc à l'État, le gouvernement propose également d'ajouter des exceptions à la transparence pour éviter de certaines publications, donc je ne reviens pas dans le détail, on lui a déjà fait aux références nous pour notre part, nous demandons des informations basiques sur les prestations de conseil qui ne sont pas couverts par le secret d'affaires comme le résumé des prestations et leur montant et ces informations devraient d'ailleurs être déjà publié au regard des règles de la commande publique, elle recoupe l'Élysée de prestation, publié par la commission d'enquête, qui n'ont soulevé aucune difficulté, en conclusion, le gouvernement ne peut donc pas se cacher derrière le secret d'affaires pour refuser de publier les informations cela serait, nous semble-t-il, juridiquement infondée et démocratiquement contestable. Oui merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, qu'on se mes chers collègues, concernant cet article 3 et par ailleurs je n'ai pas encore fait, mais je m'en soucie complètement à tous les collègues à tous les collègues qui sont intervenues précédemment pour rendre hommage à ce travail de grande qualité, de la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques plus public ce travail qui aboutit à la présente proposition de loi nos collègues Éliane Assassi et Arnaud Bazin, cet article 3, préconise la création d'un document budgétaire qui recense les prestations de conseil par les administrations publiques, englobant l'état les établissements publics, les hôpitaux sous je crois que ça a été largement développé par les collègues, on a fait les les travaux de la commission d'enquête ont mis en évidence les difficultés y compris notamment pour eux, l'état de chiffrer l'étendue du recours aux prestations de conseils avec des sommes importantes qui sont indiqués dans le rapport, sommes importantes en augmentation qui atteignent environ 900 millions d'euros, chiffre de 2021 qui ont été rappelés par différents intervenants. Donc, cet article 3 concerne donc la création d'un document budgétaire annexé à la loi de finances, qui est appelé jaune budgétaire, la notion de transparence meilleure lisibilité des des mesure approuvée par par la commission mais redéfini pour respecter le domaine exclusif des lois de finances référence également à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, donc concernant cet article 3 je me rallierait bien entendu à la vie de leurs porteurs et des collègues de la commission des lois, qui se sont investis sur ces sujets, je vous remercie. Nous avons sur cet article un amendement l'amendement trois du coup trente-deux pardon du gouvernement qui a la parole. Oui, monsieur le président, par souci de cohérence et pour que le débat puisse avancer au rythme souhaitable à cette heure tardive, je propose de présenter à la fois l'amendement 33 34 et 35 du gouvernement qui porte sur les articles 3 4 et 8 la proposition de loi je dis par cohérence puisque effectivement la proposition que je souhaite vous soumettre : c'est de fusionner ces articles là. Je vais faire en 2 temps je faire rapidement, d'abord vous dire quelles sont les réserves que j'ai que je ressens en lisant le texte tel qu'il est écrit et dans un 2ème temps, conformément à ce que j'ai dit lors de la discussion générale, je ferais la proposition du gouvernement qui je veux insister sur ce point n'est en aucun cas une proposition qui affaiblit le texte mais qui a vocation, de mon point de vue de ceux du gouvernement, à le rendre plus opérant plus efficace, efficace et au final effectif d'abord je crois effectivement que la dispersion des informations voulues par la représentation nationale dans différents documents n'est pas de nature à rendre les choses plus effectif, on aura des informations dans un rapport au Parlement jaune budgétaire, on aura des informations dans le document social unique, on aura des informations publiées au fil de l'eau, dont d'ailleurs là le le le réceptacle n'est pas très bien définie dans la loi sur les bons de commande et puis on aura un autre rapport au Parlement remis sur la question des compétences, je ne crois pas que la dispersion de ces informations dans différents rapports dans différentes temporalités soit de nature à renforcer l'effectivité de ce que vous voulez suivre au fond en tant que représentation nationale, un mot sur un de ces objets qui me sont pas convenir par rapport à l'objectif qui est voulu, c'est le document social unique, je crois que ce document social unique ce rapport social unique, ça n'est pas son n'objet l'objet du rapport social unique, il est défini par la loi et les défini même très précisément par la loi, par décret, autour de 10 rubrique l'emploi le recrutement parcours : formation, rémunération santé-sécurité au travail, organisation du travail, qualité de vie au travail : action et protection sociale dialogue social discipline je prends. Deux secondes pour citer son objet, pour bien montrer que, à mon sens, ça n'est pas l'objet d'y faire figurer l'ensemble des prestations de conseil, c'est un document qui est d'ailleurs rédigé par les RH des ministères qui n'est pas rédigé par les agents administratifs qui aurait la charge de regarder les prestations de conseil, donc je veux vraiment soulever votre attention sur ce point parce que je crois que ce serait un dévoiement de cet objet ce rapport social unique qui est bien utile, notamment dans les lignes directrices de gestion je mentionnais un point supplémentaire qui sont les temporalités diverses qui serait publié dans les différentes informations donc on aurait un rapport annuel qui serait une annexe budgétaire on aurait un rapport qui lui sera fait tous les 5 ans sur la question des compétences et puis on aurait au fil de l'eau, la publication de l'intégralité des bons de commande, là aussi, je crois que ça n'est pas de nature à rendre effective utilisable au fond cette matière ce qui est je crois la finalité recherchée dans le texte, un dernier mot sur la publication des bons de commande de façon moi je suis effectivement réservé sur ce point, non pas pour affaiblir les mesures de transparence, je vais faire des propositions nettes et précises sur cette question là, mais je crois qu'il faut regarder de façon précise opérationnel ce que serait la publication effective de tous ces bons de commande, il y a eu en 2021, 4854 commandes, le travail, je crois que vous ne remettait pas en cause, de bis-Phase, un certain nombre d'informations de caviardage un certain nombre d'informations, le nom, par exemple, des agents publics, c'est un travail qui prend du temps, Obama à peu près cinq heures par prestation de conseil, ça voudrait dire qu'on consacrerait 25000 heures de travail, je crois qu'il faut en être conscient, pour pouvoir simplement publié l'intégralité des bons de commande, là aussi, je crois qu'il y a une question de proportionnalité qui n'est pas celle recherchées par la loi, un dernier point dans les éléments, moi qui me paraissent pas convenir dans la loi telle qu'elle est écrite c'est un point qui pourrait mettre en cause la responsabilité des agents qui aurait mener ce travail de caviardage de préparation des bons de commande, ça pourrait inclure leur responsabilité devant la loi, si il commettait une erreur sur ce travail ah monumental, je crois qu'on peut en convenir qu'il leur serait demandé et donc quelle est la proposition que le gouvernement fait de faire figurer l'ensemble des informations utiles dans un document unique, donc j'ai pris l'engagement à la tribune tout à l'heure d'en faire un document qui soit gravé dans le marbre et qu'il devienne une annexe permanente de nos textes budgétaires qui soit à la disposition des assemblées chaque année porterait les informations suivantes : la publication de l'intégralité des commandes de l'État intitulé de la commande, ministère qui le commande montant ça serait des informations qui serait exhaustive qui donnerait la stratégie menée, ministère par ministère, pour contrôler le recours aux prestations de conseil, telle qu'elle est publiée, peut-être de façon imparfaite dans ce 1er document qui aura vocation à être enrichi et qui enfin qui enfin viendra préciser les transferts de compétences et donc la stratégie de réinternalisation de compétences qui sera opéré je m'arrête une seconde sur ce point parce que oui, je crois qu'il est essentiel, vous avez raison de le souligner, je crois même que c'est l'enjeu essentiel de ce texte, quels sont les moyens que se donne l'État pour réinternalisation certain nombre de compétences, je dirais qu'il y a 3 étages dans cette fusée d'abord les compétences qu'on réinternalisation de la DTP j'ai annoncé la création de 15 postes, je pense, je compte continuer cet effort de réinternalisation ensuite, c'est la mobilisation de fonctionnaires tout à fait capable, vous l'avez mentionné les uns et les autres et donc le travail mené avec ta dièse de formation de fonctionnaires bien on vous en donnerai la visibilité après année après année et enfin la mobilisation de nos corps d'inspection, parce que je suis d'accord avec ce que vous avez dit parfois, il peut y avoir des redondances entre des missions menées par des cabinets de conseil et le travail mené par des corps d'inspection, donc l'ensemble de ces informations sur l'Internet, le centre de compétences, je prends ici l'engagement qu'on les fasse figurer dans ce jaune budgétaire, un dernier mot Madame la présentation aussi parce que vous l'avez mentionné oui j'assume le fait qu'il puisse y avoir des exceptions à la publication de telle ou telle bon de commande, non pas simplement pour des questions de secret des affaires, mais je vais vous donner un ou 2 exemples très précis pour vraiment faire réfléchir l'Assemblée sur ce que nous nous apprêtons à publier, il peut y avoir des exceptions, par exemple quand le Fisc travaille à l'optimisation de la lutte contre la fraude fiscale, en s'appuyant sur un cabinet de conseil spécialiste en Intelligence artificielle, hé bien j'espère convaincre les députés, les sénateurs pardon communiste que à ce moment-là, hé bien oui j'assume qu'on ne fasse pas publicité de la stratégie d'optimisation de la lutte contre la fraude fiscale et je prends un exemple qui n'est pas un exemple théorique puisque vous savez qu'une mission a été menée pour mieux traquer notamment mieux repérer les piscines et les propriétaires de piscines en s'appuyant effectivement sur des cabinets de conseils pour mener ce type de mission, je prends un autre exemple qui je crois est illustratif de ce que nous pouvons aussi préserver, il y a parfois des cabinets de conseil qui nous aide à travailler sur des stratégies, par exemple, la stratégie hydrogène de la France, qui est un sujet sur lequel nous sommes notre pays en compétition avec d'autres pays, ben moi j'assume de dire que je ne sais pas à livre ouvert à des puissances étrangères l'intégralité du bon de commande et des missions et des intitulé que nous livre blanc et donc le principe, puisque je vous l'ai dit, je ne resterai jamais sans contre-proposition le principe dans ce jaune budgétaire, ça serait un principe de justification par les ministères de la non publication éventuelle en donnant la raison, la nature de la raison invoquée et donc vous aurez ainsi dans ce jaune budgétaire unifier toutes les demandes, je crois qu'ils sont formulées par l'Assemblée, à travers cette proposition loi pardon, j'ai été un peu long mais cela valait argumentation pour les articles 3 5 et 8, monsieur le président. David la commission s'il vous plaît madame la rapporteure. Bien, Monsieur le Ministre, document unique pérenne, jusque-là, nous nous retrouvons cependant telle que vous le proposez avec l'amendement qui vise effectivement à réécrire l'article 3 a supprimé l'article IV et à supprimer également l'article 8 vous me permettrez tout de même de de de noter effectivement que c'est à nos yeux un appauvrissement du du du travail telle validée par par la Commission puisque la suppression par exemple de l'article 8 amènerait un document qui ne comporterait plus de cartographie des ressources humaines dont dispose le ministre. C'est en matière de conseil or justement, et cela a été rappelé, y compris par un certain nombre d'un. Intervenant à la tribune, il y en a, justement, plus que jamais besoin de plus la liste des prestations, vous venez de le dire, et c'est un choix et une, nous ne le partageons pas la liste des prestations seraient en données relatives à l'accord-cadre, auxquelles se rattachent la prestation de conseil ainsi que des données relatives au marché où l'eau et au bon de commande. Ferrand ces données participe pourtant pleinement à l'objectif de traçabilité que promeut la proposition de loi vous permettez également avec la rédaction de de pardon de l'article 3 d'accroître les réserves à la publication des données, vous venez de le dire, sur la suppression de dollars. Article IV, vous me permettrez de faire un parallélisme avec la présentation commune des 3 amendements du gouvernement et donc là aussi d'émettre un avis. Un peu plus global, ce qui nous on nous fera gagner du temps par la suite sur la suppression de l'article IV simplement bien évidemment sera la villa aussi défavorable mais la publication ordonnée ouvert des informations relatives aux aux prestations de conseil des bons de commande constituerait l'aboutissement, à nos yeux, du mouvement de transparence et d'ailleurs, je souhaite rappeler à cette occasion que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique l'prévoit que l'ouverture des données publiques et la règle et que la mise à disposition des données de référence ont une facilité leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'État sur la suppression de l'article 8. J'y suis déjà je suis déjà intervenu, donc je n'y reviens pas et donc, vous l'aurez compris, ce sera un avis défavorable sur ces trois amendements.

je suis suivrai pas le gouvernement sur ces, sur ces 3 articles, je voudrais rappeler notamment qu'en matière de fraude fiscale, on a eu et qu'énormément de difficultés à obtenir, notamment sur la fraude à la TVA, le moindre conseil extérieur alors qu'on nous a expliqué en long, en large et en Technicolor que les ressources internes étaient suffisantes, total, on est le dernier

pour le logiciel Louvois, dont on sait que ça a été un succès foudroyant, donc moi je me fie au travail de notre commission d'enquête et je ne voterai pas les amendements du gouvernement. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, merci de vos explications, vous avez donné 2 exemples assez précis et c'est bien de pouvoir donner des exemples, je pense qu'en matière de stratégie industrielle, des questions se posent. Sincèrement, vous avez évoqué la question de l'hydrogène, je pense que la question spatiale, la question des télécommunications, la question énergétique, bon ça voudrait un débat au Parlement, qu'on puisse regarder quelles filières industrielles, il nous faut protéger d'intérêts étrangers, par contre vous donner, hein, le 1er, exemple, pardonnez-moi, ça nous fait sourire ici sur ces mômes sur l'évasion fiscale, ce qu'on veut bien savoir quel cabinet nous aide et aide le ministère de l'Économie et des finances sur la question, l'évasion fiscale, espérons que ça ne soit pas McKinsey parce qu'autrement, il pourrait se mettent sur les premiers sur la liste, puisque eux-mêmes pratiquent l'optimisation fiscale plein pot non, voilà, il faut, il faut nous dire : ben oui, pardonnez-nous, mais lorsqu'on ne paye pas d'impôts pendant 10 ans, il y a une il y a une question donc : on veut bien savoir le cabinet qui nous aide pour savoir si au moins, eux, sont en adéquation sur la question fiscale, voyez donc on entend bien le 2ème argument qu'on peut mettre en débat avec avec ici le Parlement sur le premier comme notre collègue Madame Goulet on pense quand même que c'est une questions régaliennes et que il faut qu'on ait des fonctionnaires suffisamment nombreuses et nombreux pour pouvoir effectuer cette mission et sur ces bancs, nous n'avons cessé de vous dire que la réduction du nombre de personnel sur précisément cette question, la fraude fiscale et l'optimisation fiscale n'est pas simple mais qu'elle mérite un certain nombre de fonctionnaires pour pouvoir faire véritablement leur travail, d'autant plus que la fraude fiscale, pèse lourdement évidemment dans le déficit de l'État, voilà je vous remercie, monsieur le président. Chemise. Sénateur, vous avez vu, je suis très respectueux de la proposition de loi et j'essaie vraiment d'argumenter, mais mes mes positions en donnant des exemples concrets, je vous avoue que ça n'empêche pas. Parfois avec un peu de malice, de bien choisir ces exemples là et j'ai, j'ai choisi un exemple qui je savais vous ferai réagir sur un sujet auquel je vous sais évidemment attachés et croyez-le c'est bien partagé, et si la lutte contre la fraude fiscale je ai pas pris un exemple en l'air, en l'occurrence, j'ai pris un vrai projet qui a abouti, qui a même donné lieu à des articles dans la presse sur la capacité pour le Fisc à mieux traquer ceux qui mènent des fraudes et notamment les possesseurs de piscines, c'est un projet qui a été menée avec l'appui de mon administration et la plus d'un cabinet, donc je voulais simplement ici vous rassurer en vous indiquant que ce n'était pas McKinsey, si telle était le sens de votre question mais oui je réitère cette affirmation dès lors que le principe de non-publication de l'intitulé de la commande de son montant et du ministère et justifiée, je sais bien, la proposition que je fais ce soir dans le jaune budgétaire, ainsi d'ailleurs Madame la rapporteure que l'intégralité la question des compétences, donc ça n'est pas enlever du Champ, ça serait bien intégré dans ce document budgétaire unique qui serait portée à votre analyse : dès lors que ce principe est justifiée, je crois sincèrement pas que ça soit un recul et on peut assumer et c'est effectivement un bon débat et vous avez eu l'amabilité de citer les sujets industriels sur lequel on peut avoir ce débat là mais ça donnerait justement la bonne prise pour expliquer que sur tel ou tel sujet il y a des travaux, mais que nous ne souhaitons pas publier ou des bons de commande ou même des intitulés de comment. Oui, sur la traque des piscines non déclarés, c'est quand même savoureux cet exemple Monsieur le Ministre, excusez-moi de rebondir Google devait 7 milliards à la France, ils ont transigé 1 milliard je crois qu'nous on fait un chèque, on a discuté et on a transigé effectivement aujourd'hui Google en remerciement, entre guillemets, va aider le gouvernement à repérer les piscines non déclarés, je ferme la parenthèse, ça devient complètement cocasse 2ème question est-ce que vous êtes prêt, Monsieur le ministre a publié le rapport que McKinsey a produit sur le métier d'enseignant qui a été cité à de nombreuses reprises dans des échanges dans le rapport est-ce que vous allez rendre ce rapport public. Monsieur le ministre. qui nécessite beaucoup beaucoup de travail, de la part de chacune des administrations qui est coordonné par le secrétaire un général du gouvernement pour pouvoir publier, ministère par ministère, l'intégralité des documents, le ministère de la transformation et de la fonction publique à communiquer l'intégralité des commandes qui étaient demandés par les journalistes concernés à la Cada et ce travail là se poursuit et l'intégralité des documents qui ont été demandées, avec un avis favorable de la Cada seront effectivement transmis aux journalistes qui les ont demandé. Bien je. Peut mettre aux voix, il y a plus de demandes de parole je mets aux voix l'amendement 32 du gouvernement qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission. Qui est favorable qui vote pour. Contre n'est pas adopté. Donc nous en revenons au texte de l'article 3 que je mets aux voix qui est pour.

Il y a pas de demande d'expression, donc je le mets aux voix, c'est le même vote. Qui est pour. Contre, faire adopter. Du coup, nous avons l'article 4 dans son état naturel, si j'ose dire que je mets aux voix qui est pour. Contre il était adopté. à l'article 5, nous avons un autre amendement 43 présenté par le gouvernement. Je le présente brièvement, Monsieur le Président, parce que je veux dire ici que je partage la finalité de l'article 5 qui est de mettre fin aux missions pro Bono, donc ça soit dit extrêmement clairement exactement pour les raisons que vous avez indiqué, je propose de modifications à ces articles, une qui est d'écriture, si je puis dire, pour venir préciser la mention que vous avez vous-même porté à l'article 238 bis, ça c'est vraiment un amendement de de pure légistique et puis sur les sujets d'écriture pour permettre la réalisation à titre gracieux de prestations de conseil entre administrations la rédaction actuelle du texte ne le permettait pas et donc rendez par exemple impossible la réalisation d'une mission gratuite par. Une université au bénéfice d'une administration et donc j'ai proposé de lever cette exception et puis 2ème point que je propose de porter, c'est d'établir une seule exception à l'interdiction d'émission pro Bono sur les situations les plus exceptionnel qu'on a rédigé à dessein dans des termes extrêmement en disant : en cas de circonstances exceptionnelles complément tant la vie ou la santé de la population, une guerre ou une pandémie, pourquoi, parce qu'on peut comprendre que dans ces moments-là, il y a des temps d'urgence qui ne correspondent pas tout le temps au temps des démarches administratives, par exemple, pour pouvoir passer des commandes, et donc c'est la seule exception que je soumets à la mise à enfin des prestations pro Bono par des prestataires privés. Madame le rapporteur. de conseil réalisateur à titre gratuit puisque il me semble que si l'article 5 ne précise pas explicitement que les prestataires et les consultants sont visées par des interdictions posées le Champ d'. Question de la proposition de loi est défini à l'article 1er que donc, dès lors, on peut déduire de cet article 1er que l'interdiction des prestations de conseil, réalisé à titre gratuit, vaut pour les prestataires et les consultants. Sur le 2ème point. Que vous venez d'évoquer Monsieur le Ministre, sur la dérogation proposée en cas de circonstances avec son compromettant la vie ou la santé de la population, bon, tout d'abord, il existe aujourd'hui dans les règles de la commande publique qu'un acheteur peut passer un marché public sans publicité. Ni mise en concurrence, près à la Hallab lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu'il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Et surtout, il revient et nous l'avons vécu il y a peu, peut encore, il revient à des éventuels, loi d'urgence qui inévitablement seraient prises. Dès lors que nous sommes dans des circonstances qui compromettent la vie ou la santé de la population, il revient aux éventuelles, loi d'urgence de revenir si besoin sur ce principe général d'interdiction, donc nous ne nous ne sommes pas pardon pour une inscription en tant que telle dans la loi, je vous remercie. Je mets aux voix l'amendement 41 proposée par le gouvernement et faisant l'objet d'un avis défavorable de la commission. 43 pardon. Qui est pour.

parfaitement rédigés en y ajoutant fait point très particulier qui consiste à interdire aux prestataires ou consultant de fournir des prestations de conseil à un client qui a bénéficié de mécénat de leur part dans les 5 années qui précèdent a fait prévenir et d'empêcher, en fait, l'instrumentalisation volontaire à un moment donné du mécénat à des fins commerciales, de façon à préparer un contrat voilà. Madame le rapporteur. Oui, il nous sommes que déjà à l'article 5 et 11 de la. Proposition de loi à constitue un cadre à la fois solide et équilibré pour les prestations de conseil réalisés au titre du mécénat, nous ne voyons pas de raison particulière encadrer davantage encore les prestations de conseil réalisés au titre du mécénat comme vous me proposer mes chers collègues, et donc nous émettons un avis défavorable. Je soumets au vote l'amendement 17 avec l'avis défavorable de la commission et le même avis du gouvernement, qui est pour.

monsieur le président je voulais préciser que l'amendement précédent avait été établi avec une association qui s'appelle Sherpa qui travaille beaucoup sur ce sujet le l'c'est l'amendement numéro en fait c'est c'est un amendement additionnel qui a pour but, en fait de préciser le le recours aux prestataires consultant privé pour la rédaction des études d'impact et la rédaction d'exposer de motifs de projet de loi est interdit, nous pensons effectivement ça a été dit, je crois, à d'autres moments de ce débat que cette rédaction doit être exclusivement réalisés par les services de l'État autre autre chose pour éviter toute dépossession du rôle de l'État et des politiques en matière d'orientation de politique publique, je citerai juste un seul l'exemple pour pour aller brièvement en 2018 le gouvernement d'Édouard Philippe, avait décidé de lancer un appel d'offres pour sous-traiter à une entreprise, l'exposé des motifs à l'étude d'impact de sa future loi sur les transports. Tu pourrais quand même un peu surprenant pour moyennant 30000 euros hors taxes, ça avait un peu alerter l'opinion publique sur les problèmes d'externalisation fait des processus de rédaction de loi donc, nous souhaitons apporter cette précision Avis de la commission. devant la représentation nationale. Cela étant, je souhaite d'abord rappeler que le grand 3 de l'article 2 de cette PPL crée en l'état une obligation de transparence quant à la participation de cabinets de conseil à la rédaction de documents pour le compte de l'administration, ce qui inclut, bien évidemment, les études d'impact les exposés des motifs des projets de loi et donc cette obligation. De transparence devrait assurément, j'ai envie de dire freiner cette partie qui a été fortement réprouvé, comme vous le disiez oh mon cher collègue, y compris qui a pu heurter aussi un certain nombre de nous. Concitoyens je, je, je crois, là pour le coup, qu'un certain nombre comme comme déjà précédemment de de mesures sont prises se suffisent à elles-mêmes et que cet amendement serait superfétatoire et insister peut-être sur la capacité à. Voir dans l'effectivité de cette proposition de loi qui, comme je le dis en entraînera finalement tout, tout le monde a à travailler et à agir différemment, je n'en doute pas, je voudrais prendre un exemple un peu parallèle au débat que nous avons ce soir mais la remarque que vient de faire notre collègue Bernard Roche précédemment pour préciser que l'amendement précédent avait été travailler avec l'association Sherpa, je crois que pour un certain nombre, nous pouvons dire il y a ici une dizaine d'années, bien peu d'amendements dans l'exposé même de leur motif précisé avec quelle association qui est l'organisme les amendements avaient pu être rédigé été déposée par nos collègues, ça devient de plus en plus monnaie courante à travers un certain nombre d'amendements déposés ici de de tous les groupes d'ailleurs et de toutes origines, preuve en est, je crois que parfois il y a la loi il y a la volonté et puis ensuite il y a une pratique qui devient monnaie courante, et je crois que c'est ainsi en tout cas que nous devons peut être rassurés en l'état, j'émettrai un avis défavorable. Oui vous avez raison madame la rapporteure, c'est la vérité qui vous rendra libre pour reprend des citations bibliques du questeur sur. Simplement pour dire que j'ai la même opinion que la rapporteure ce ce point et cet amendement, ça me permet simplement de souligner que le gouvernement était pleinement favorable aux mesures qui ont été portées dans les premiers articles et notamment à la fin de ce que je qualifierais des marques blanches, c'est-à-dire des situations, on ne sait pas qui tient le crayon est-ce que c'est le cabinet de conseil est-ce que c'est le cabinet du ministre est-ce que c'est une administration et, donc, cette avancée-là est pleinement soutenue sans aucune réserve par le gouvernement et je pense qu'elle répond en grande partie à l'amendement qui est proposée, donc même avec rapporteur. mais j'essaie de réfléchir à cette question de l'étude d'impact, s'agissant de l'exposé des motifs, vous avez 1000 fois raison, il suffit que le ministre-l'écrive mais alors pour l'étude d'impact, nous avons déposé une proposition de loi avec monsieur Montaugé là-dessus parce que je ne sais pas s'il vous arrive de lire les études d'impact moi je dois vous dire que c'est quelque chose de très ennuyeux, on a envie de s'endormir quand on lit cela pourquoi parce que l'étude d'impact est faite par les services du Ministre qui présente la loi, donc là, forcément, c'est l'État. Mais alors, aucun ministre ne va publier une étude d'impact qui critiquera son projet de loi, c'est-à-dire que les services du ministère disent que l'impact de la loi est très bon. En général, ce qui fait que cette littérature un peu compassé n'est pas intéressante et je suis d'accord que ce n'est pas forcément à McKinsey ou autre, qu'il faut confier l'étude d'impact, moi je ferais plutôt confiance à des organismes scientifiques, par exemple, des universités, le CNRS, l'INSERM, enfin un certain nombre de d'organismes qui ne serait pas dans l'optique de dire forcément du bien ce que feront les fonctionnaires du ministère, qu'on je pense qu'il faut réfléchir à cette question parce que je crois que les études d'impact tels que sont aujourd'hui sont une fausse bonne idée. C'est quand même une obligation constitutionnelle,

Donc il n'est pas adopté. à l'article 6 H, la parole est à Madame Müller Bronn. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'ai souhaité prendre la parole sur cet article car il constitue un pilier essentiel de la proposition de loi pour mettre fin à l'opacité dont le gouvernement fait preuve aujourd'hui encore, en effet, le document tant attendu par le Sénat et obtenu début octobre sur le détail des missions et leurs prix laisse perplexe les dépenses, ils sont toujours très élevés puisque leur coût total dépassera en 2022, son niveau d'avant la crise sanitaire, environ 230 millions d'euros ce coup nous interroge sur le maintien de certaines missions dont le caractère superflu, voire inutile, avait été pourtant largement documentés, tant par le Sénat, que par les enquêtes journalistiques, enfin le contenu du document restent trop évasifs pour contrôler les et les objectifs de ces prestations, à titre d'exemple, on apprend que l'entreprise italienne techno homme Biette a réalisé 6 missions pour le ministère de la transition écologique, d'un montant de 25,3 millions d'euros, il s'agit, selon le document d'études géophysiques pour l'implantation d'un parc éolien au large de la Bretagne, on lit que le prestataire a mis à disposition un navire et un équipage pour étudier les zones d'implantation, réaliser des tests de forage en pleine mer, etc le etc semble un peu léger pour comprend des justifier une dépense de plus de 25 millions, vous en conviendrez, c'est pourquoi il faut impérativement inscrire dans la loi le contenu, l'évaluation et les conséquences concrètes de des prestations fournies merci. Merci l'amendement 35 présenté par le gouvernement sur l'article 6. Oui, monsieur le président, là aussi pour soutenir pleinement la finalité de l'article 6 qui est de renforcer le principe d'évaluation des prestations de conseil. Je suis d'ailleurs remarquer que ce principe là il était inscrit dans la circulaire du 19 janvier 2022 par le 1er ministre qui en prenaient effectivement l'engagement et c'est un principe qui a été intégrée dans l'accord-cadre renouvelé la DTP que j'ai eu l'occasion de présenter tout à l'heure avec d'ailleurs un modèle type établi par la DTP que je tiens à votre disposition pour encadrer pour normer au fond la façon dont on évalue les prestations de conseil donc soutien total à la finalité d'articles, un amendement qui porte sur 2 modifications qui sont au fond des mises en cohérence la première mise en cohérence, c'est avec le débat que nous devons que nous venons d'avoir sur les secrets protégés par la loi, c'est simplement de la cohérence complète, je refais pas le débat ici mais je pense que c'est cohérent de le porter sur les sujets d'évaluation de la même façon que nous n'avons porté sur la publication des missions de conseil la 2ème mise en cohérence, c'est une mise en cohérence avec la loi de 1978 qui s'était penchée justement sur les documents publiés par les administrations et qui avait donné un article L 311 de du code des relations entre le public et l'administration qui justement disait que les évaluations ne devaient être publiés que pour des décisions qui étaient prises par l'autorité et par la puissance publique et donc ça mettait une exception qui était déjà prévu dans la loi de 78 sur les évaluations sur des décisions ou des avis n'était pas encore pris et rendu par l'État, notamment par le gouvernement pour une prise de décision dans la sérénité et donc je propose au Sénat de se mettre et de garder la conformité et la vie du législateur de 1978 sur cette question là.

oui à travers effectivement cet amendement le le gouvernement cherche à exclure l'obligation de publication, les évaluations des prestations de conseil qui portera atteinte à l'ensemble des secrets protégés des secrets protégés par la loi, ainsi que les évaluations qui porterait sur les prestations de conseil préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration d'élaboration, pardon, excusez-moi, la rédaction de de de cet amendement semble certainement un peu trop large en ce qu'elle englobe notamment le secret des affaires qu'elle risque d'avoir pour conséquence de priver d'effectivité, une grande partie des dispositions prévues à l'article 6 qui existe déjà un certain nombre de protection, notamment sur les décisions administratives ont. Pour, je pense que c'est un vrai sujet en tout. Qui, qui qui est proposé en l'état, ce sera un avis défavorable, mais avec la volonté en tout cas de réfléchir et de trouver une rédaction qui répondent aussi quand même à un certain nombre d'impératifs qui pourraient nécessiter des protections. Simplement d'un mot parce que sur la la mise en cohérence avec la loi 78 je trouve que c'est vraiment dommage, et en l'occurrence, affaiblir la loi de de ne pas intégrer cette modification là j'en profite pour pour apporter une précision supplémentaire, c'est dès lors que la décision publique a été rendue et prise cette exception à la non publication de l'évaluation tombe d'un évidemment et l'évaluation et publié de façon plaignants. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, en introduisant subrepticement le secret des affaires qui jusque-là ne figure pas dans le texte fou ajouter quelque chose qui peut être très lourde de conséquences et qui peut faire exploser tout l'intérêt du texte parce que, y compris les cabinets de conseil pourront exciper à tout moment du secret des affaires, et je crains beaucoup que ce que vous nous proposez là soit quelque peu déflagration heure par rapport à l'exigence de transparence qui est la nôtre. Je soumets au Sénat, l'amendement 35 proposée par le gouvernement avec l'avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre, il est pas adopté, du coup je mais aux voix, l'article 6 qui est pour. Contre il est adopté, je mets aux voix, l'article 7. Monsieur. suis saisi l'opportunité, monsieur le président de l'explication de vote pour préciser un petit peu les choses et et les éclaircir et puis je voudrais bien, en fait vous entendent, Monsieur le Ministre, sur cet article et savoir ce que vous en pensez, sur le fond, bon en France, il y a pas de police, de la langue, voilà déjà faut faut démystifier tout ça ne ne pas être dans la caricature dans le privé, sur les réseaux sociaux, les gens entre eux ils parlent bien comme ils veulent, il y a pas de difficulté de ce côté-là et encore heureux, et puis plus on rentre dans les interactions sociales comme c'est pas le monde du travail plus règle apparaissent et se précise ici de quoi parle-t-on, on parle des pouvoirs publics, on est bien dans ce couloir-là, c'est-à-dire que le chef de l'administration, le 1er ministre et puis les les ministres avec lui sont là pour faire appliquer un droit qui découle un certain nombre de normes la constitution : la loi Toubon ensuite par exemple les circulaires, je prends l'exemple des circulaires primo-ministériel quand on dit qu'on féminise les titres Madame la préfète, par exemple, ben c'est comme ça et pas autrement et s'il y a des préfets dans certains départements, qui continue de se faire appeler Madame le préfet, elles sont en contradiction avec ce que disent leur administration, de la même façon, quand Édouard Philippe, par circulaire précise les choses sur la question uniquement du point médian est pas de l'écriture inclusive de tous les fantasmes qui vont avec, de tous côtés, d'ailleurs, il n'en a parfaitement le droit, il demande simplement à son administration de s'exprimer d'une manière qui soit clair et pas d'une autre, donc ce que nous entendons par là à travers cet article, c'est en fait, faire en sorte de saisir une opportunité de faire en sorte que la loi Toubon soit précisé pour qu'on sache que non seulement l'administration a l'obligation de travailler en français de s'exprimer en français, mais qu'en plus elle que, elle doit exiger de ce qu'elle paye pour lui rendre des documents qu'il en fasse autant, donc on ne pourra pas étendre ces dispositions par exemple aux grandes entreprises, y compris quand elles sont issues de grands monopoles d'État, qu'elles ont, qu'elles ont une belle histoire publique je pense notamment à la Poste, qui arrivent à pondre des, des, des, des idées aussi idiote que Ma French Bank, malheureusement on ne peut pas aller sur ce genre de de dispositions ça viendra peut-être un jour mais c'est pas le bon véhicule législatif pour le faire et en tout cas, on en reste vraiment à ce que l'administration s'exprime en français, il restera une question qui est celle de la bonne application et ça, ça relève quasiment uniquement de de l'administration et de ceux qui dirigent, administration et là-dessus, mais vous pourrez compter sur le Parlement pour contrôler cette bonne application mais je suis curieux de savoir ce que vous pensez, sur le fond de cette disposition. Monsieur le Ministre, répondez à la. Sollicitation aimable de Monsieur et j'ai, j'ai fait observer au Sénat que en une heure 3 quarts, nous avons fait la moitié du travail. Alors, je ferai preuve de sobriété dans ma réponse pour vous dire que je suis tout à fait favorable à cet article-là, et j'en profite pour saluer le travail de la commission des lois et de son président qui a donné une accroche en l'intégrant et en faisant référence à la loi Toubon ce qui je pense lui donne une base solide.

comme la présidente à Cécile a dit en fait, dans son intervention lors de la discussion générale, l'article 2 de la Constitution prévoit déjà que le français est la langue de la République, donc il me semble que cet article est déjà satisfait et je je dirais même plus parce que c'est peut-être c'est avant la révolution donc sais ce que que Madame Assassi là oublié, mais en fait en France l'édit de Villers-Cotterets de 139 est toujours d'application et il précise très clairement 1539 la langue de l'administration française et le français et ne peut pas être une autre langue, à l'époque le concurrence latin, maintenant c'est l'anglais, que je suis pas contre le principe que c'est déjà satisfait comme nous on ne veut pas des lois bavardes, c'était peut-être inutile. Je mets aux voix, l'article 7 qui est pour.

monsieur Benalla, Roche, il a la parole. Oui, Monsieur le Président, cet amendement dix-huit a pour objet de préciser que dans le rapport présenté au Parlement, le Conseil supérieur de la fonction publique, dont il est question dans cet article le libellé des postes occupés et les compétences attaché aux fiches de postes des fonctionnaires soit précisé, il est également demandé au gouvernement de motiver dans ce présent rapport les recours qu'il peut faire prestataire ou un consultant externe comprenait bien le but, définir les postes permettent de savoir avec chaque poste, quelles sont les compétences nécessaires et ensuite voir pour quel usage, le gouvernement va faire appel à des prestataires en fonction justement de ses compétences et des postes qui sont occupés.

n'est pas adopté, du coup, je mets aux voix, l'article 8. Pas l'intervention qui est pour l'article 8. Il est donc adopté je mais aussi aux voix, l'article 9 je ne fait pas l'objet de demandes de parole. Qui est pour.

qui concerne les obligations déontologiques des cabinets de conseil, et des consultants, comme je l'ai dit, lors de la discussion générale, nous assistons depuis quelques années, un renforcement des règles dans toutes les sphères de la société, et tant mieux. Je vous rappelle une citation du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, devant la commission d'enquête le 26 janvier dernier, je cite, l'intervention des cabinets de conseil peut légitimement susciter des inquiétudes en matière de déontologie ces risques, nous les avons documenté avec la commission d'enquête et ils ne sont pas virtuels, ce matin même le journal Le Monde publiait un article sur le risque de conflit d'intérêt dans la gestion du plan de relance européen, l'État a le droit et même le devoir, de connaître les autres clients de ces cabinets de conseil qui ne doivent pas pouvoir servir 2 intérêts divergents en même temps, c'est pourquoi nous sommes très circonspects face aussi prochains amendements qui seront présentés par Monsieur le Ministre, en matière de déontologie les reculs souhaitée par le gouvernement sont en effet nombreux reculs sur le périmètre des déclarations d'intérêts qui ne concernerait plus que les dirigeants des cabinets de conseil recul sur les moyens de contrôle de la Haute autorité qui ne pourraient plus faire de contrôles sur place, alors que la majorité des autorités indépendantes le peuvent recul sur la saisine de la Haute autorité pour la transparence par les représentants des fonctionnaires recul sur les amendes administratives qui seraient remplacées par des sanctions pénales, beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre, chacun le sait, recul sur le contrôle du pantouflage lorsqu'un consultant intègre l'administration et réciproquement et enfin recul sur les modalités d'entrée en vigueur, vous ne souhaitez pas que notre PPL et des effets rétroactifs ce qui voudrait dire que les nouvelles règles ne s'appliquerait ni à l'accord-cadre de l'UGAP, concluait l'été dernier, ni à l'accord-cadre de la TP qui sera conclu en fin d'année, j'ose espérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que cela ne reflète pas la volonté du gouvernement, vous comprendrez donc Monsieur le Ministre, que nous ne pourrons être favorable à vos prochains amendements la navette permettra d'améliorer encore le texte, mais nous souhaitons nous ne souhaitons pas, pardon pas revoir son ambition à la baisse, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les conflits d'intérêts. Donc nous avons examiné l'article l'amendement 36 proposée par le gouvernement qui va le présenter. Merci monsieur le président, d'abord je voudrais indiquer ici que le renforcement de la déontologie et une finalité du texte qui est aussi recherché par le gouvernement, je profite pour dire le soutien, j'ai pas pris la parole pour pas faire perdre autant d'un débat sur l'article 9 que nous venons d'adopter et qui entraîne des renforcements déontologique pour le texte, je fais aussi remarquer que, et dans la circulaire du Premier Ministre du 19 janvier 2000 22 et dans l'accord-cadre renouvelé la DTP nous avons intégré des mesures renforçant le contrôle déontologique et notamment les déclarations sur l'honneur des consultants sur lequel je vais revenir mon point porte sur ses déclarations, des consultants à la fois sur des questions de proportionnalité et d'effectivité des finalités qui sont recherchés par la loi, la proportionnalité d'abord ce qui est voulu ici, c'est d'avoir une publication exhaustive. Pour l'ensemble des consultants, je fais remarquer ici que le terme de consultants entraînerait nécessairement et probablement une appréciation sur l'ensemble des salariés, des cabinets de conseil, il y a à peu près 120000 salariés dans les cabinets de conseil en à 15 % qui travaille avec l'État et donc cela voudrait dire qu'on aurait des dizaines de milliers de personnes concernées par des déclarations d'intérêts exhaustive pour eux et pour leurs conjoints exactement les mêmes qui sont demander à des parlementaires ou à des ministres, que nous sommes, ça veut dire que le moindre consultant qui arrive dans un cabinet de conseil qui démarre en tant que junior sur une mission, il est soumis exactement une déclaration exhaustive, ainsi que sa conjointe ou son conjoint, son son concubin sur ses activités professionnelles, j'ai ajoute j'en profite pour le faire, je le referais pas sur l'article 12 que vous y avez ajouté en commission une possibilité. De contrôle sur place par la HATVP, qui n'est même pas existantes pour vous ou pour moi en tant que parlementaire, en tant que c'est-à-dire que je, je, je, j'insiste sur cet argument de proportionnalité par la loi telle qu'elle est rédigée, aujourd'hui vous faites peser sur des consultants juniors, voire même sur des employés, des cabinets de conseil des dispositions qui sont plus exigeantes que celle que nous nous appliquons en tant que parlementaire, ou en tant que ministre, je crois effectivement qu'il y a des vrais sujets de proportionnalité, j'insiste sur le risque constitutionnel que représente la rédaction de l'article, en l'état je crois très sincèrement qu'il ne passerait pas et fourches caudines du Conseil constitutionnel, il y a déjà eu cette question qui a été posée lors de l'examen pour la transparence de la vie publique, le Conseil constitue c'est a estimé que le recours élargi à une telle obligation de déclaration pour les conjoints entraîner une atteinte disproportionnée au droit constitutionnellement garanti à la préservation de la vie privée, ça ce ce, pour des questions de proportionnalité j'essaie vraiment très sincèrement de vous convaincre de la bonne foi du gouvernement sur ces questions-là, j'insiste sur le sujet de l'effectivité, quel serait le résultat concret de la loi telle qu'elle est portée aujourd'hui, nous aurons donc probablement des dizaines de millions. Pardon, des dizaines de milliers, c'est déjà suffisant de déclaration exhaustive d'intérêts qui seraient fournis aux administrations non pas aux référent déontologue des administrations, mais probablement aux acheteurs dans les administrations qu'leur arriverait entre leurs mains quand fera-t-il quelles seraient les possibilités de prise en charge par les administrations de ces dizaines de millions de déclarations exhaustif d'intérêt qu'ils leur arriveraient je crois que nous aurions un réel problème d'effectivité et qui d'ailleurs pourrait mettre en danger, y compris la responsabilité des agents publics parce que si il y avait un conflit d'intérêt effective par la suite, on dirait : mais vous avez eu entre les mains, cette déclaration d'intérêt qu'on avait vous fait et il s'agit là d'un acheteur quelqu'un qui est pas comme la HATVP, spécialisé dans l'analyse des déclarations d'intérêt sauf à penser que vous voulez que l'intégralité des déclarations d'intérêts remontent à la HATVP et je pense qu'on aurait un problème d'embolisation de la HATVP, donc j'ai des vraies réserves sincère effective sur la rédaction, cet amendement, je reste là non plus pas sans contre-proposition je propose et le gouvernement propose de centrer les déclarations exhaustive d'intérêt sur les dirigeants, ainsi que sur les cabinets de conseil qui, par là même répondrait à la question que vous avez posée, vous avez dit à juste titre, on veut connaître les autres clients des cabinets de conseil, la rédaction telle que proposée par le gouvernement permettrait de le faire et donc sans tronc les déclarations exhaustif d'intérêt sur les dirigeants et sur les cabinets de conseil et demandons pour le coup à l'exhaustivité des consultants de fournir mission par mission, une déclaration sur l'honneur de non conflit d'intérêts sur la mission sur lequel ils auraient à intervenir, document, j'insiste sur ce dernier point qui serait opposable juridiquement et pénalement opposable c'est un conflit d'intérêts étaient avérés et donc je crois que la proposition que je fais n'est pas du tout un affaiblissement en matière de déontologie mais au contraire une proposition pour rendre plus effectives, la finalité de la loi telle que vous la portée. Si Monsieur le Ministre, madame la rapporteure. Oui, ce sera un avis défavorable et je m'en remettrai par gain de temps aux éléments apportés par le président bassin peut être 2, juste Monsieur le Ministre pour pour préciser sur les éléments que vous avez donnés puisque, effectivement, le Conseil constitutionnel, tout d'abord, censure sur l'élargissement aux parents et aux enfants, et là, cela est circonscrit uniquement aux conjoints

la la Haute autorité. Que donc il n'y aura pas une comment une remise en question. De de de la vie privée, comme cela semble être une grande inquiétude, hein, puisque les cabinets de conseil. Eux-mêmes le disent : moi je voudrais simplement dire : je sais que j'ai donné déjà plusieurs fois cet exemple là, vous savez, moi je me souviens des débats que nous avons eu ici au moment de la mise en place de la loi de la transparence et les débats que nous avions, y compris dans les couloirs et dans les pièces annexes où tout nous avions tous eu très très peur de tous les bancs d'ailleurs de ce que ça allait engendrer en matière de débat allemand de la vie privée des uns et des autres, je garderai pour le sucré des murs toutes les blagues et boutade qui ont pu être dites en dehors de cet hémicycle pour autant aujourd'hui finalement certes ce cela peut être vécu parfois comme une contrainte, les élus dans leur très grande majorité s'y plie, il y a un caractère public il y a un caractère consultables dans les dans les préfectures, à la demande des citoyens, il y aurait certaines odeurs des choses à Rome peut être plus perfectible mais finalement, cela se fait-il, on ne commande pas, y compris à chaque publication pour telle ou telle Ministre pas dans la presse, la vie des uns et des autres, donc je crois qu'il faut pouvoir rassurer et c'est finalement en généralisant la transparence que nous la désacralise on peut être et rassureront ceux qui en seront pour l'instant, jugés comme les victimes mais que demain je pense, nous aiderons. monsieur le président, chemise, juste un mot rapide, nous ne demandons pas la publication de la déclaration d'intérêts du conjoint, on demande juste qu'il soit précisé sa profession et d'ailleurs c'est ce que vous avez fait vous-même dans le cas de l'accord-cadre de la DTP, donc ça doit pas soulever de difficultés particulières, mais on a besoin de savoir, en effet, pour les gens qui interviennent, quelles sont leurs propres intérêts, d'autre part, l'acheteur, qui va éventuellement être destinataire de cette déclaration d'intérêt s'il ne s'estiment pas suffisamment armés pour en juger, je pense que les cas seront quand même pas très nombreux, bien il pourra se retourner vers la HATVP ça été prévu donc, c'est pourquoi nous souhaitons maintenir le dispositif telle que nous l'avons proposé. Je mets aux voix l'amendement 36 du gouvernement avec cet avis défavorable de la commission qui est pour. Contrôle.

Et on n'a pas été adopté. à l'article 11 nous avons l'amendement numéro 22 présentée par Madame Duranton. Merci Monsieur le Président, cet amendement a pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d'État prix a pris après avis public de la H pardon, excusez-moi, VP la définition des modalités de publication des informations relatives aux actions de démarchage de prospection et de mécénat le dispositif que nous vous proposons d'adopter s'inspire de celui prévu par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Et l'avis de la commission va l'avoir porteur. Défavorable, monsieur le président. Monsieur le Ministre. Il y avait favorable Monsieur le présent en insistant simplement sur un point, c'est que ce décret sera rendu après avis public comme l'a indiqué à la sénatrice Duranton, de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et donc il y aura bien un avis donner un travail mené avec la Haute autorité pour rédiger le décret d'application de cette. Oui. monsieur le président, Monsieur le Ministre, nous avons confiance dans le gouvernement mais la prise d'un décret présente toujours un risque pour rappeler un souvenir un peu délicat, le président de la HATVP évoque souvent les représentants d'intérêts et la loi Sapin II, qui est bien écrite, nous rappelle-t-il, mais il souligne aussi le fait que le décret qui a été pris en application là complètement dévitalisé le poids, le problème persiste depuis maintenant plus de 5 ans, donc si on pouvait éviter de reproduire les mêmes erreurs, ce serait très bien. je mets aux voix l'amendement 22 de notre collègue Nicole Duranton, qui est pour.

aucune organisation syndicale ne peut saisir une autorité administrative indépendante, ça serait un précédent absolu que nous créons, à travers la proposition de loi, je ne crois pas que ce soit le rôle des représentants syndicats et j'ai un respect absolu pour les organisations syndicales que de saisir. La Haute autorité sur les sujets des cabinets de conseil, le rôle des organisations syndicales, c'est de protéger les agents de la fonction publique, en l'occurrence c'est de représenter leurs droits et leur intérêt et je crois qu'on viendrait dévoyé le rôle des organisations syndicales, en proposant une telle possibilité de saisine 2ème sujet : je l'ai déjà évoqué donc je serai très bref sur le rôle et le pouvoir donné à la Haute autorité de contrôle sur place pour l'ensemble des salariés, des cabinets de conseil encore une fois, nous créons là un précédent et je crois une inégalité devant la loi, que, en l'occurrence je, je, avec laquelle je ne suis pas du tout du tout à l'aise en donnant ce pouvoir de contrôle sur place sur l'ensemble des salariés qui n'existe même pas, ni pour les ministres, ni pour les parlementaires. Madame l'apporter. L'avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement 37 présenté par le gouvernement, qui fait l'objet d'un avis défavorable de la commission qui est pour.

il y a un refus suite à une demande de communication de pièces ou de documents par la Haute autorité, transparence de la vie publique dans ce cas, il est proposé que la Haute autorité saisisse la commission des sanctions qui est mise en oeuvre à cette fin, notamment et je tiens à remercier particulièrement Madame Cécile Cukierman qui a fait des propositions très judicieuse, de manière à ce que cet amendement, qui était un parfait soit meilleur. Ah, de la commission favorable, Monsieur le Ministre. Défavorable par cohérence avec les positions que j'ai porté par ailleurs sur l'examen du texte. Pas l'intervention donc je soumet au vote du Sénat, l'amendement 25 avec avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement. Qui est pour.

pour. Il est adopté à l'article 13 il y a un amendement trente-huit du gouvernement, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le président, et de la même façon que j'ai pu le faire précédemment, je propose de de porter les amendements sur les articles 13 14 et voir 15 puisque il me semble, formé au fond un un un lot cohérent, si je puis dire, au fond le débat que nous avons là, à travers ces amendements dépasse à mon sens le périmètre de la. Son doigt telle qu'elle est étudiée, c'est le rôle même de la HATVP, ça renvoie à des débats sur la loi de transparence ou sur la loi sapin qui avait été porté à l'époque sur le rôle et le pouvoir que nous donnions à la Haute autorité de transparence pour la vie publique et je crois en effet que nous remettre ont fondamentalement en cause la façon dont a été pensé la Haute autorité si nous adoptions les articles tels qui sont portés pour les cas spécifiques, des cabinets de conseil se porte effectivement sur les régimes de sanctions, il s'avère que le législateur s'était déjà penché sur ces questions et le bon régime de sanctions applicables sur les représentants d'intérêts, en l'occurrence il avait admis une exception sur les contrôles sur place, exception qui avaient été données à la Haute à la Haute autorité de pouvoir faire des contrôles sur place chez les représentants d'intérêts, mais en l'occurrence, malgré cette exception avait été réaffirmée un pouvoir de sanction qui était un prof sanctions pénales et qu'il n'était donc pas un pouvoir de sanction, porté par la HATVP de pouvoir de sanction administrative, donc il me semble qu'il serait effectivement une dissonance par rapport au rôle de la HATVP au droit telle qu'il ait pensé aujourd'hui par le législateur de créer ce pouvoir de sanction spécifique pour les seuls, cabinet de conseil, après on peut avoir un débat sur qu'est-ce qui est le plus dissuasif, moi je crois que les sanctions pénales, telle que définie par la loi sont des sanctions qui sont en réalité dissuasive, j'entends parfois que la HATVP serait, au fond, démunis de ce pouvoir de sanction et que son rôle serait du coup inopérant, ça n'est pas vrai, la HATVP a déjà transmis des éléments au procureur de la République, un bon nombre de fois pour être très précis, il y a 178 dossiers qui ont été transmis par la HATVP à la justice depuis 2014 il y a eu 28 condamnation condamnation effective et définitive sur des ministres sur des parlementaires, c'est quelque chose qui est totalement effectif aujourd'hui et donc, je crois, c'est un dispositif qui n'est pas du tout inopérant au contraire qui me semble être largement dissuasif l'article 14 ben je porte un amendement de suppression qui est très largement cohérent avec ce que je viens d'indiquer, parce que je suis contre la création d'un régime de sanctions, donc d'une commission qui lui est liée et puis sur l'article 15 je crois effectivement que ce sont aussi des amendements de cohérence de cohérence avec le droit aux aux Européens le dispositif de sanction pénale prévoit aussi des mécanismes d'exclusion des marchés publics et des mises en cohérence avec le droit européen sur des mécanismes déjà existants d'auto apurement qui sont prévues par les textes européens et donc c'est pour ça que je souhaitais vous présenter l'ensemble de ces amendements d'un bloc, si je puis dire. Entendu alors sur l'amendement trente-huit l'avis Oui, merci Monsieur le Président, je pense qu'en 2 minutes, je ferais également un un Tir groupé, si vous me le permettez, ce sera un avis bien évidemment défavorable parce que, au contraire, nous pensons, et ce n'est pas qu'une effectivement une question de procédure mais que la sanction administrait administrative sera en la matière bien plus efficace. Parce que plus rapide dans son dans son application par rapport à une sanction pénale qui prend beaucoup plus de temps, nous sommes donc demeureront favorable à la création d'une commission des sanctions et par rapport à ce que vous évoquiez, monsieur le Ministre, oui, parce qu'il y a qu'un particulier cas spécifique à travers cette question des cabinets de conseil et je crois que depuis le début, vous le voyez bien l'objectif n'est pas de de généraliser à d'autres champs mais de garder le le le le définition initiale de cette proposition de loi, il y a besoin de, de, de, de, de commissions qui peuvent ne pas exister dans d'autres cas, et donc d'où la volonté de maintenir la création de cette commission des sanctions au sein de la Haute autorité et par voie de conséquence, à ce que je viens de dire, sur l'article 13 et 14 l'amendement numéro 15 est également défavorable, toutefois je je tiens tout de même à préciser que, dans le respect du droit européen, la proposition de loi à l'article 15 prévoit justement un mécanisme de régulation, en s'appuyant sur une collaboration, je cite, active qui reprend la la disposition de la directive entre la Haute autorité, d'une part et l'administration qui a bénéficié de la prestation de conseil donc pour ces raisons, ce sera des habits d'ores et déjà défavorable sur ces trois amendements présentés par le gouvernement. Madame Assassi Madame Assassi d'abord. Merci Monsieur le Président, simplement un mot pour aller dans le sens de madame la rapporteure et simplement rajouter que l'amendement du gouvernement telle qu'il est rédigé en fait supprime des sanctions par exemple lorsqu'un cabinet de conseil réalise une prestation pro Bono ou le logo de l'administration, ce que, ce qui pour nous est inacceptable bien évidemment. Donc je mets aux voix l'amendement trente-huit du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est favorable, qui est pour. Qui est contre. Ah, l'abstention, il est donc repoussé et un amendement 31 de Madame Goulet, qui va nous le présenter. Oui, monsieur le président, Monsieur le ministre, on peut dire. Il est rédactionnel, il s'agit de remplacer total par consolider. Oui c'est un avis défavorable parce que rédactionnel mais peut-être pas compris non plus que défavorable, je vous demanderai un retrait puisqu'avec l'expression totale puisque consolider nous. Nous en parlions se déforme avec ce qui est déjà loi dans l'article 20 autant de la loi de 78 pour la CNIL, mais c'est également ce qui est utilisé pour définir le montant de la sanction pécuniaires qui peuvent être prononcées par l'Autorité des marchés financiers qui là aussi par le chiffre d'affaires annuel total ah rédactionnelle quand même qui nous met en difficulté, c'est plus une demande de retrait hein madame monsieur bonjour, tiens voilà. Du coup, je mets aux voix, l'article 13 lui-même qui est pour.

nous avons un avis défavorable de la commission, je suppose que le vote du Sénat est le même que sur les amendements précédents, il est donc écarté et donc je soumets au Sénat l'article quatorze, qui est pour.

Oui, monsieur le président de l'examen attentif. Des dispositions qui visent à entraîner l'exclusion de la commande publique omettent d'Indy de viser l'article 434 13 du code pénal qui est celui du faux témoignage l'histoire et l'expérience de cette commission d'enquête nous montre que ce genre de choses peut arriver donc il s'agit de d'ajouter : Alice, des infractions qui peuvent entraîner l'exclusion de la commande publique, les personnes qui auraient été condamné pour ce motif. Monsieur Bouquet. Oui, même esprit pour notre amendement, je vais rappeler l'un des temps forts de cette commission d'enquête qui fait le Buzz comme on dit aujourd'hui on bon français excusez-moi chers collègues qui, qui a fait beaucoup parler, voilà et on se souvient de cette affirmation de Monsieur Teste, j'ai dit une qui était à l'époque, ex-directeur associé du cabinet McKinsey, qui a dit : je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France mais le président Bazin a rappelé tout heure les pouvoirs d'investigation, d'une commission d'enquête et c'est très bien ainsi, et la commission d'enquête s'est rendu sur place à Bercy et s'est rendu compte que McKinsey n'avait pas payé d'impôt sur les sociétés sur au moins 10 ans alors que le chiffre d'affaires de la firme en France atteint 329 millions d'euros en 2020 par exemple, dont environ 5 % d'ailleurs réalisé dans le secteur public et qu'il y emploie environ 600 salariés, un phénomène de parjure à l'évidence, puisque ça a été rappelé les les propos sont tenus, sous serment, et donc ce qui a valu de saisir le bureau du Sénat qui a invoqué l'article 40 de du code de procédure pénale pour suspicion de faux témoignage, ça n'est pas rien donc nous estimons à l'instar de notre collègue Nathalie, vous voulez que, pas question de donner le moindre Euro d'argent public à un cabinet qui serait con de enfin convaincu de parjure dans ce genre de situation et donc interdiction de soumissionner un quelconque marché public, voilà le sens de l'amendement que nous proposons. Et l'avis de la commission madame la rapporteure. Un mot pour dire que mon cabinet qui n'a eu besoin d'aucun cabinet de conseil pour me donner cette position m'indique qu'il aurait certainement des difficultés d'écriture par rapport à la conformité aux textes européens mais ce que je vous propose, c'est dans l'esprit très constructif de pouvoir travailler à l'occasion de la navette, l'écriture de cet amendement, si on peut l'améliorer, donc avis de sagesse du gouvernement sur cet amendement dont je partage la finalité. Je soumets. Au Sénat, donc les deux amendements 9 et 46. Avec l'avis favorable de la commission et la sagesse du gouvernement qui est pour.

15 l'article car le l'amendement quarante du gouvernement qui l'a présenté, si je me souviens bien. Qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission s'il n'y a pas de demandes de paroles je soumet au vote. De l'assemblée, c'est le même vote. Il est donc repoussé quant à l'article 15, lui-même, je le mets aux voix qui est pour. Et contre il était adopté. Sur l'article 16, nous avons l'amendement 41 du gouvernement. Oui, monsieur le président, sur la question du contrôle des aller-retours entre le public et le privé qui est le dernier débat que nous aurons au fond sur sur ce que je note, c'est que la rédaction de l'article s'écartent très nettement de la loi de transformation de 2000 et des principes qui avait été introduit. Non pas par le gouvernement à l'époque, mais par le Parlement à l'époque sur l'architecture de contrôle déontologique dont la HATVP dit le plus grand bien, et mécanismes de contrôle que se sont appropriés les administrations cet article au fond de distorsion par rapport au mécanisme dans la loi de transformation premières distorsions en considérant que il n'y a plus aucune hiérarchie dans les agents concernés, c'est-à-dire que ça concernerait, contrairement à ce que dit la loi de transformation qui était centré sur les postes à responsabilité au sein des administrations qui me semble-t-il et l'exercice et l'objectif et la finalité visée par le texte de loi de pouvoir éviter les influences la première distorsion absolument tous les agents administratifs sont concernés par le dispositif, telle que vous l'avez créé, c'est-à-dire un agent administratif, tout en bas de l'échelle hiérarchique aurait les mêmes prérogatives ou le aura les mêmes contraintes en termes de contrôle par la HATVP que les postes à plus fortes responsabilités premières distorsions 2ème distorsion vous créez un régime ad-hoc pour les cabinets de conseil, je peux en comprendre la philosophie mais donc, on a une distorsion qu'il considérerait que, au fond, il y a moins d'enjeux déontologiques moins dangereux d'influence pour un haut fonctionnaire qui représenterait, qui rejoindrait, par exemple, l'industrie de l'armement et qui viendrait du ministère des Armées que pour un simple fonctionnaire très bas dans l'échelle hiérarchique qui rejoindrait un cabinet de conseil pour diversifier son parcours professionnel, donc je crois là aussi que dans une logique de proportionnalité et d'effectivité du texte, il vaudrait mieux se reposer sur l'architecture, créé par la loi de transformation qui vise à ce que les responsables de l'administration puissent d'abord regarder c'est une situation de conflit puisse en référer au référent déontologue et en cas de difficultés remonter à la HATVP pour les postes concernés, je pense que c'est un mécanisme qui a fait ses preuves, qui fonctionne et sur lequel nous devrions pouvoir nous reposer. Oui, peut-être, sans surprise, mais ce sera un avis effectivement défavorable, vous me permettrez, non pas par l'heure tardive, parce que j'avais prévu de vous le dire en tous les cas, mais de dire peut-être que c'était un compromis un peu bancal que que vous proposez, monsieur le Ministre, puisque d'un côté on tente dopé, entre le droit commun et la dérogation qui est visée à l'article 16, j'aurais envie de dire tout simplement soit effectivement le sait. Lors du Conseil rentre déjà dans le cadre des dispositions prévues aux différents articles cités du code général de la fonction publique et donc dans ce cas là, bah allons jusqu'au bout et supprimons cet article 16, soit au contraire, et c'est la position en tout cas, qui a été celle de la commission, il est nécessaire effectivement de premières dispositions spécifiques pour l'activité de conseil privés et même si j'entends les réserves que vous avez mise nous souhaitons en tout cas les laisser en l'état, de, de, de, dans la rédaction de cet article et donc de gagner en tout cas en clarté et lisibilité je vous remercie des favoris. Monsieur le Ministre. Un mot sur la prestation bancal que que que vous mentionnez, en l'occurrence elle part de l'intention d'améliorer le dispositif actuel de l'architecture dans la loi de 2019 en mentionnant les enjeux spécifiques liés au cabinet de conseil et en s'appuyant sur la HATVP pour leur demander de nous aider dans la rédaction des lignes directrices de gestion justement pour mieux travailler avec les référents déontologue dans les administrations et donc, au contraire, c'est un mécanisme je crois tout à fait effectif et améliorer que je viens la proposer.

d'ailleurs, on le rappelle, dans l'exposé des motifs, ce qui qui restera bien le périmètre, il semblerait que dans le texte de l'article, on ait parlé d'agents publics, c'est vrai qu'il peut y avoir à ce moment-là, une difficulté, je crois que dans la navette, ça pourra être améliorée précisé en tout cas ce que nous visons sont les responsables publics et pas tous les agents publics clairement ensuite on en a évalué le nombre dans les précédentes années, c'est un nombre assez limité de personnes qui va se compter en un peu plus d'une centaine à l'année, la transmission à la Haute autorité ne présente pas de difficulté, je pense, d'examen et on a évolué à ce sur ce sujet, une véritable zone de risque, j'ai donné un exemple tout à l'heure, un responsable de cabinet de conseil qui prend un poste à l'Élysée, qui fait venir ce cabinet de conseil pour rien réorganiser le service, donc il a la responsabilité, ça c'est une vraie zone de risques, on a besoin de d'avoir délimité tout ça par une transmission à à la vie de la HATVP pour qu'elle fasse des exclusions nécessaire par la suite et qu'elle se donne les moyens du contrôle, ça nous paraît tout à fait proportionnée, pour le coup est réalisable. Dernier mot pour pour indiquer quand même que le rapport de la commission des là des lois pardon mentionne aussi la mention agent public, donc je crois que très sincèrement l'Arctique telle qu'il est aujourd'hui n'est pas bien rédigé et concernerait l'ensemble des agents publics, donc je crois qu'il a quand même un vrai problème de rédaction qui est là et vous mentionnez un cas particulier de recrutement par l'Élysée d'un cas qui je crois n'aurait pas été remis en cause par la HATVP, et sur lequel aucun conflit d'intérêt ensuite n'a été mentionnée sur le cas particulier que que vous visez, donc je crois que le dispositif, telle que prévue par la loi, en l'occurrence c'est un un cas particulier on, on, on avait échangé, en amont de ce texte ne aurait pas été visés par le dispositif proposé, j'ai l'occasion de le vérifier. Je mets aux voix l'article l'amendement 41 présenté par le gouvernement avec l'avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre, il n'est pas adopté quant à l'article seize je le soumet au vote qui est pour. Contre, il est donc adopté. Je se met également au vote du Sénat, l'article 17 qui ne fait pas l'objet d'amendement qui est pour. Qui est contre pas l'abstention, il était adopté, à l'article nous avons un amendement numéro 23 de Madame Durand ton et de ses collègues. qui nécessite un haut niveau de sécurité des systèmes d'information, nous souhaitons ainsi assurer la compatibilité de l'article dix-huit avec les directives européennes relatives à la passation des concessions et des marchés publics qui prévoit que les exigences en matière de recevabilité et de sélection des candidatures ne sont destinées qu'à garantir qu'un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière, ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat.

les audits en sécurité informatique, qui sont exigés, où donc, c'est pour cette raison que j'émets un avis favorable. Je mets aux voix l'amendement ainsi discuter le numéro 23 avec un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il y a pas d'abstention, il n'est donc repoussé, nous pouvons donc voter sur l'article 18 qui est pour.

Oui, c'est tout simplement d'un moment de suppression de l'article 19 pour une raison extrêmement simple, c'est que l'article 19 ne me paraît pas conforme au droit régissant la relation contractuelle et l'article 2 du code civil indiquant que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif votre assemblée avait eu à examiner en 2017 le le le le projet de loi ratifiant l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, vous aviez à l'époque, réaffirmer la protection constitutionnelle des contrats en cours, je pense que vous la remettrai en cause en adoptant l'article 19 telle que rédigée. Oui, ce sera un avis défavorable et nous savions, j'ai envie de dire des pointes de début, il y a, il y a un véritable débat le le souhait en tout cas telle qu'il a été retenu et que la proposition de loi s'applique notamment aux accord-cadre de l'UGAP et de la DTP qui vient d'être renouvelé récemment en ce qui concerne l'UGAP ou qui fait l'objet d'ailleurs d'un d'un d'un d'une procédure de renouvellement actuel pour l'accord des TP, je crois que ces accords-cadres, nous le savons et d'où peut être aussi, c'est cette volonté à travers cet article 19 représentent des sommes significatives qui ne peuvent être ignorés. Le le montant du nouvel accord-cadre de la TIPP de la DTP pardon, estime à 150 millions d'euros hors taxes pour la période 2023 2027 avec un plafond à 200 millions d'euros, ils sont donc excessif d'attendre que ces accords-cadres expire dans 4 ans pour que la proposition de loi puisse s'appliquer enfin et pleinement et donc en outre l'absence d'application immédiate, impliquant la modification des accords-cadres aurait pour conséquence une rupture d'égalité entre les prestations de conseil se rattachant un accord-cadre et celle contractée en dehors de ceux-ci pour toutes ces raisons, un avis défavorable.

donc l'amendement est repoussé et j'voir l'article 19 qui est pour. Qui est contre il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, y a-t-il des demandes d'explications de vote Madame Duranton. au nom du groupe RDPI je souhaite saluer la qualité de nos débats, je me réjouis de constater que l'objectif poursuivi par la proposition de loi est largement partagée sur les bancs de notre assemblée, les modifications apportées au texte initial, vont dans le bon sens, à commencer par celles relatives au Champ d'application parmi les autres avancées figurent l'interdiction pour l'administration d'attribuer une adresse électronique au consultant je mentionnerait également l'obligation pour les prestataires de conseils de produire les conclusions d'un audit attestant d'un niveau minimal de sécurité pour ce qui concerne les mécanismes de transparence et de contrôle déontologique des ajustements sont nécessaires pour ne pas dire indispensable aussi nous regrettons que nos amendements n'ait pas été adoptés nous regrettons également que l'Euro également le rejet des amendements présentés par le gouvernement, à l'instar du ministre et nous souhaitons que la proposition de loi chemine, nous sommes en effet convaincu que la navette permettra de trouver un point d'équilibre, et donc d'aboutir à un dispositif effectif et proportionnée, la navette sera aussi l'occasion de trancher la question des modalités d'inclusion des collectivités territoriales dans un Champ d'application, vous l'avez dit madame la rapporteure le débat de ce soir est un point d'étape et non un un un aboutissement pour toutes ces raisons, les groupes RDPI votera pour la proposition de loi. Ensuite Madame Goulet. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, très brièvement, compte tenu de, de leur avancée pour dire la, la, la satisfaction qu'on peut ressentir, après le travail qui a été fait, non seulement pendant la commission mais aussi

pour rendre ce ce texte de meilleur et et plus précis, un regret toutefois, c'est de ne pas avoir voté l'amendement numéro 11 d'autres collègues Bénard Roche qui, qui proposait d'interdire les les prestations pour la rédaction d'étude d'impact et d'exposé des motifs d'une loi, je pense que ce sujet est vraiment extrêmement important qu'il s'agit là d'une délégation de ce qu'il y a de plus régalien dans nos ministères, c'est-à-dire l'arrêt la la rédaction de propositions de loi, les études d'impact, je vois bien ce que ce qu'a voulu dire notre collègue sueur, ça peut porter à discussion, mais franchement l'exposé des motifs et les textes, sachant que les cabinets d'avocats, n'offre strictement aucune garantie sur les Liens d'intérêt pour ne pas dire les conflits d'intérêts, je pense que ce sujet-là sera vraiment à creuser durant la navette et ça me semble aussi extrêmement important, donc nous nous reverrons sur ces sujets, nous nous reverrons aussi sur le PLF dans quelques jours pour un jaune ou un orange budgétaire sur les sujets dont nous avons parlé ce soir donc, nous voterons évidemment avec enthousiasme le texte qui a été débattu ce soir. Ensuite, monsieur Bazin. Oui, merci Monsieur le Président, ce Ministre pour vous dire simplement que le groupe Les Républicains votera le texte tel qu'il est sorti de nos débats ce soir ce soir rebondir quand même un instant sur ce que disait Madame Goulet sur l'amendement proposé par Monsieur Bénard Rochon, étude d'impact, moi on m'indique à moi qui ne suis pas du tout juriste, mais qui aura une difficulté parce que cela relèverait d'une loi organique, donc ça fait, c'est un exemple pour dire qu'il y a un certain nombre de choses encore à regarder, on en est bien d'accord dans les détails pour parfaire et cette proposition de loi la navette est là pour ça et et nous lui faisons confiance le principal, c'est que l'esprit de l'architecture de la proposition de loi ont été conservées Qui serait aveugle en matière de déontologie serait en danger, je l'ai dit tout à l'heure et je crois que quand tous ces dispositions là seront bien stabilisé auront été définitivement adopté, vous verrez Monsieur le Ministre, que toutes les administrations sont porteront mieux parce qu'elles seront sécurisés dans leurs rapports avec cabinet de consultants et de même les ministres pourront aussi être plus serein et plus tranquille, je pense qu'on a fait un travail intéressant vraiment sur le fond, totalement transpartisan, on a encore une fois, conserver l'esprit et les objectifs de cette proposition de loi, c'est pourquoi nous le voterons avec beaucoup de satisfaction. Je vais mettre aux voix la proposition de loi et j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains sur l'ensemble du texte ben donc être procéder au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56.

Plus personne ne demande à voter Le scrutin est donc clos. Résultat du scrutin votants 344 exprimés 331 pour le projet de la proposition de loi 331 contre 0 la proposition est donc adopté. Hé, chers collègues, j'avais levé la séance prochaine séance, mercredi 19 octobre c'est-à-dire aujourd'hui à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement, la séance est levée.